La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il constitue un pan essentiel de notre pacte social fondé sur la solidarité entre tous, sans distinction de catégorie professionnelle ou de génération. C'est à juste titre que nos compatriotes y sont très attachés. Pourtant, on ne peut ignorer les changements profonds qui touchent notre pays : le vieillissement de la population, la diminution du ratio entre actifs et retraités, ou encore des déficits budgétaires difficilement soutenables. Ne rien faire serait irresponsable, alors que les incertitudes minent notre cohésion nationale. Nos concitoyens le savent bien, eux qui attendent aujourd'hui de l'équité,

Cette réforme doit intégrer non seulement les projections démographiques de long terme, mais aussi les transformations des modes de vie qui découlent de l'allongement de l'espérance de vie. Non, les seules considérations budgétaires ne constituent pas un dogme

Nous nous réjouissons, en particulier, que le Parlement soit associé à la définition de la valeur du point. Il appartient désormais aux partenaires sociaux de débattre de ce projet dans le cadre d'un dialogue social apaisé. Pour l'heure, les Français sont très attentifs, à juste titre. Monsieur le Premier ministre, qu'aucune catégorie professionnelle ne sera perdante

que notre objectif n'était pas de faire, çà et là, telle ou telle petite économie, mais de dire la vérité aux Français. Compte tenu des transformations du monde professionnel, du caractère haché

faire. Il fallait le dire clairement : c'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai fait, tout à l'heure, devant le Conseil économique, social et environnemental, quand j'ai présenté un projet de réforme

Monsieur le Premier ministre, ce midi, vous avez franchi la ligne rouge : vous êtes hors-jeu et vos annonces vont continuer à faire coaguler toutes les colères Avec votre projet de casse des retraites, les Français vont travailler plus longtemps- jusqu'à 64 ans -et toucheront des pensions plus basses. Alors que les salariés du secteur privé comme du secteur public, ainsi que les jeunes, sont massivement mobilisés depuis jeudi dernier, vous maintenez votre projet funeste d'instauration d'un système de retraite par points soumis aux aléas économiques et financiers. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez effectivement pas fait d'« annonces magiques ». En revanche, vous vous êtes lancé dans un excellent numéro de bonneteau dont personne n'est dupe Malgré l'illusion de la concertation sociale, la majorité de la population a bien compris les dangers de votre projet de réforme des retraites. Malgré vos belles promesses qu'il n'y aura ni vainqueurs ni vaincus, ceux qui vont pouvoir se frotter les mains sont les marchés financiers, à l'instar de ces financiers casseurs reçus par le Président de la République- les BlackRock -qui attireront les salariés qui en seront capables vers les retraites par capitalisation. Les lignes directrices de votre réforme n'ont pas bougé d'un iota.

sûrement mieux que le revenu de nos agriculteurs, qui attendent en vain les résultats de la loi Égalim. Vous allez sûrement mieux que nos étudiants, qui ont perdu 35 millions d'euros de crédits dans le projet sûrement mieux que nos aides-soignants, nos urgentistes, nos enseignants et nos retraités, qui ne sont pas dupes quand ils observent la progression exorbitante des rémunérations des patrons du CAC 40 et les dividendes de 50 milliards d'euros dont vous avez allégé la fiscalité. Ce ruissellement-là, celui de l'argent-roi, existe bien ! C'est vous et vous seul, monsieur le Premier ministre, qui en êtes responsable ! Dans un contexte délétère et anxiogène, terreau de la poussée de l'extrême droite dans notre pays, vous avez franchi de nouvelles lignes rouges avec les annonces que vous

et les corps intermédiaires, n'êtes-vous pas en train de briser notre contrat social, fondement de notre pacte républicain ?

C'est un point de vue que je respecte ! Sa conséquence mécanique est que, au moment où vous avez quitté les affaires, tout allait vraiment mieux

Monsieur le Premier ministre, la France est aujourd'hui divisée en deux camps : ceux qui râlent et ceux qui râlent contre ceux qui râlent ! Ces derniers jours, on a surtout entendu les premiers. Je voudrais parler des autres, de tous les autres, de ceux qui ne défilent pas, de ceux qui n'ont ni mégaphones ni pancartes, parce qu'ils savent qu'un examen objectif des faits est toujours trop long pour une banderole, et de ceux qui ne font pas grève et se font parfois à ce titre injurier ou crever leurs pneus. ceux qui ne supportent plus de voir que, lorsqu'on a un problème avec le Gouvernement, on s'en prend aux travailleurs naufragés dans des transports à l'arrêt, aux enfants se heurtant à des grilles d'écoles fermées, aux chefs de petites entreprises ... Je vois que les râleurs ne sont pas seulement dans la rue aux chefs de petites entreprises, disais-je, supportant seuls le coût de l'absentéisme forcé de leurs employés, aux commerçants qui espéraient rattraper les pertes subies l'an dernier, mais voient s'annoncer pour Noël de nouvelles pertes, pour le plus grand profit d'Amazon ! Je veux parler de ceux à qui l'on dit que le service public a une obligation de continuité, mais qui constatent que 90 % des grèves ont lieu dans le secteur public, ceux qui remarquent que les soi-disant défenseurs du service public s'en prennent en priorité aux usagers de ce même service et que le baratin de la grève au service de tous n'est que le faux-nez de la défense de privilèges corporatistes. Ces Français-là sont beaucoup plus nombreux que les grévistes. Néanmoins, comme ils ne manifestent pas, personne ne se soucie d'eux ; ils continuent donc de ramer en attendant un métro qui ne viendra jamais ou un train qui sera supprimé. Comme si cela ne suffisait pas, la CGT nous annonce désormais le blocage des raffineries. Bonjour, les fêtes de Noël en famille ! Bonjour, la démagogie ! Nicolas Sarkozy avait réussi, en 2007, à faire adopter une loi sur le service minimum qui a fonctionné pendant quelques années. Elle est désormais bafouée et inopérante. Ma question est la suivante, monsieur le Premier ministre Premier ministre : pouvez-vous nous assurer de la détermination du Gouvernement face aux blocages présents et annoncés ? N'est-il pas temps, comme le proposent certains de nos collègues, de réfléchir à de nouvelles dispositions sur le service minimum garanti ?

avec votre style inimitable et d'ailleurs inimité, vous décrivez une réalité préoccupante.

les dénoncent ; ce que je regrette, c'est que le choix des uns puisse passer par la dénonciation Nous vivons dans une démocratie ; nous devons donc assumer nos choix et nos positions. Ceux qui font grève en ont le droit, mais ils doivent le faire conformément à la loi.

des films ! Ces pressions ne sont évidemment pas acceptables. De la même façon, tous les mouvements qui consistent à nier

qui s'incarne dans un régime universel de retraite est exactement porteuse de la logique inverse, selon laquelle tous les Français, quel que soit leur statut, quel que soit leur métier, contribuent à la retraite de tous les Français.

ou de production. C'est illégal ; nous faisons donc intervenir les forces de l'ordre pour que ces blocages ne puissent prévaloir ! Cela n'est pas toujours facile, car nous savons très bien quel risque

Nous avons bien compris que le retour à l'équilibre du système actuel serait l'affaire des partenaires sociaux et que l'âge pivot serait fixé à 64 ans d'ici à 2027, et non 2025, mais vous n'avez rien dit, monsieur le Premier ministre, du coût des mesures de transition et des mesures nouvelles ni de la manière dont vous allez les financer. La parole

et annoncées, nous ne nous payons pas de mots et nous assumons nos responsabilités. C'est à ce prix que nous pourrons construire un système universel équitable et responsable.

posées. Le Gouvernement a déjà abandonné l'objectif d'un retour à l'équilibre des comptes publics en 2022. Alors, où allons-nous dans les cinq ans qui suivent ?

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je vous propose de parler d'un autre sujet : le commerce international. En octobre dernier, le président Trump a annoncé plus de 7 milliards de dollars de taxes punitives sur les produits européens. Cette annonce intervenait après le feu vert de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'institution ayant évalué les dommages pour les États-Unis du fait des subventions accordées à Airbus par l'Union européenne. Il s'agissait de la plus lourde sanction jamais imposée par l'OMC,

Ces taxations punitives à répétition risquent d'affecter durablement l'économie mondiale et mettent déjà en difficulté un grand nombre des entreprises françaises. Les producteurs de vins français estiment le préjudice à plus de 250 millions d'euros par an et ils craignent un effondrement global de leur activité : d'abord des pertes de ventes, puis, plus grave, des pertes de marché par déréférencement.

que répondez-vous aux professionnels qui font aujourd'hui les frais de ces dissensions et appellent les autorités françaises et européennes à négocier des solutions ?

qu'ils ont donnée à la France, en août, en marge du G7, à revenir à la table des négociations à l'OCDE et à accepter cette solution internationale de taxation des géants du numérique.

Aujourd'hui, à 50 ans, si l'on a changé plusieurs fois de métier, vouloir connaître le montant de sa pension s'apparente à du masochisme. À 40 ans, si l'on a subi une carrière difficile, précaire ou hachée, tenter d'estimer sa pension invite à une dépression certaine. À 30 ans, imaginer sa retraite s'apparente plus au fantasme qu'au rêve. Être une femme, c'est avoir la certitude d'une pension de retraite inférieure de 42 % à celle d'un homme. Notre système, fondé il y a plus de soixante-dix ans, est devenu au fil des réformes une jungle qui provoque l'anxiété et qui oppose les Français les uns aux autres plus qu'il ne les unit. En retrouver l'ADN ne pouvait plus passer par des réformes paramétriques. Monsieur le haut-commissaire, depuis deux ans, vous avez réalisé une large concertation, dont l'organisation a été louée par les partenaires sociaux, puis plus récemment par les Français que vous avez rencontrés au fil des réunions organisées dans l'ensemble du pays. Tout ce travail a permis au Premier ministre et au Gouvernement de proposer un nouveau cadre qui va refonder tout notre système. Il s'organise autour de quatre piliers : l'universalité au travers d'un système unique de cotisation par points ; l'équité, car chaque euro travaillé donnera les mêmes droits à chacun la gouvernance ouverte qui garantit la prise en compte de tous, la stabilité à long terme et la certitude que la valeur du point et les pensions progresseront ; la solidarité par la suppression des 42 caisses, la confortation de notre régime de répartition et la protection des familles et des plus fragiles.

Une chose est certaine, les régimes de retraite doivent être réformés. Je vous le dis d'autant plus que notre famille politique a assumé des réformes courageuses dans ce domaine. Il y a eu les réformes Balladur, Fillon, Woerth. Il faut rendre à César ce qui est à César ! Ces réformes ont sauvé de la faillite le régime de retraite de nos compatriotes, car elles ont eu le courage de toucher à la durée de cotisation, même si cela ne plaît pas à tout le monde dans

La deuxième : que devient, dans cette réforme, la majoration de trimestres dont bénéficient les mères de famille ? Est-elle supprimée ? Que devient la majoration de 10 % par parent pour les familles de trois enfants ? La troisième : que deviennent les réserves des régimes des salariés du privé ? Vous avez simplement évoqué l'avenir de celles des régimes des professions libérales. La quatrième : le bonus-malus s'appliquera-t-il dès 2022 ? Et si oui, s'appliquera-t-il aux régimes spéciaux ? La cinquième : les salariés pourront-ils, comme aujourd'hui, bénéficier d'une reconstitution de carrière complète à 67 ans ?

revanche, un certain nombre de ces réformes méritent d'être corrigées. Vous évoquez la réforme de M. Balladur : sur les 70 milliards

Nous allons rectifier cela, en indexant les points acquis sur l'évolution des salaires, ce qui est une avancée considérable, y compris pour la fonction publique. Vous évoquez la réversion. Il existe actuellement treize systèmes de réversion ! Lorsque nous avons consulté nos concitoyens ainsi que les partenaires sociaux, ils ont tous été favorables à la proposition qui consiste à garantir 70 % des ressources du couple. À quel âge ? Et nous réfléchissons

Celles-ci seront désormais calculées « en temps réel » sur la base des ressources du trimestre précédent, et non plus de celles qui auront été perçues deux ans plus tôt. Vous présentez cette réforme comme une mesure de justice. Or l'économie qu'elle va engendrer- 1,4 milliard d'euros d'après vos estimations -se fera au détriment des familles les plus modestes et des jeunes qui entrent dans la vie active. Une fois de plus, ce sont précisément ceux qui ont le plus besoin de justice sociale qui vont faire les frais de votre politique. Chacun sait que les jeunes de 18 ans à 24 ans qui démarrent leur vie professionnelle,

Et c'était précisément le principe des APL : elles permettaient de les soutenir pendant quelque temps encore, même si leur situation évoluait positivement. Depuis le début du quinquennat, les aides au logement sont la cible de votre gouvernement : baisse de 5 euros, 5 euros, suppression de l'APL accession et, aujourd'hui, réforme du mode de calcul. Depuis 2017, l'impact de ces réformes s'élève déjà à 7 milliards d'euros. Ce sont autant d'atteintes portées au pouvoir d'achat des jeunes actifs et des ménages les plus modestes. Monsieur le ministre, quelles mesures d'accompagnement avez-vous prévues prévues pour ces personnes qui vont perdre brutalement leurs APL et se retrouver dans les plus grandes difficultés

L'usage du transport public augmente dans les habitudes des Français ; c'est une réponse essentielle aux enjeux environnementaux. La fiabilité du transport public, sa continuité sont les conditions de son développement, mais surtout une exigence pour tous ceux dont c'est le seul moyen de transport. Trop souvent et en particulier depuis sept jours, la réalité est tout autre. Si le droit de grève est un principe fondamental de notre démocratie, ce que nous respectons, il est malheureusement devenu le droit de bloquer. Trouvez-vous tolérable que bus, métros, RER, TER, Transiliens soient à l'arrêt ou presque ? Des heures interminables de galère, la boule au ventre, matin et soir, sous la pluie et dans le froid, pour aller gagner leur vie et le droit de payer leurs impôts pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter à proximité de leur lieu de travail. C'est inadmissible ! Le droit de grève n'est pas le droit de bloquer le pays. Ne pensez-vous pas que ce qui est possible pour la télévision publique devrait l'être pour les transports publics ? Et

Nous sommes également sensibles à la situation de tous ceux qui ont besoin d'aller travailler et de se déplacer et qui connaissent des difficultés. La situation est actuellement la suivante : environ un tiers des Transiliens fonctionnent en Île-de-France, deux lignes de métro automatisé fonctionnent, certaines lignes

d'État, ma question était pourtant simple et elle appelait une réponse par oui ou par non ! Depuis une semaine, quelques milliers de grévistes paralysent 27 millions d'actifs. Cela coûte 400 millions d'euros par jour aux entreprises. Avez-vous conscience de l'exaspération des Français ? Les entendez-vous ?

est dans notre ADN de républicains de trouver des solutions pour ne pas aggraver davantage la situation de la France en Europe et dans le monde.

Monsieur le ministre, le 5 septembre dernier, vous annonciez un plan de lutte contre les violences subies par les sapeurs-pompiers, sans même attendre la remise des travaux conduits ici, au Sénat, par Catherine Troendlé, Patrick Kanner et moi-même sur le sujet. La mesure phare de votre plan était la mise en place de caméras-piétons. Cette mesure est bonne, mais elle n'est pas à porter à votre seul crédit. La loi prévoyant le dispositif est d'ailleurs d'origine sénatoriale- sur l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Decool -et son décret d'application était déjà pris depuis plusieurs semaines au moment de l'annonce.

où en êtes-vous de la mise en oeuvre des engagements que vous avez pris devant les sapeurs-pompiers et, surtout, comment envisagez-vous d'intégrer les propositions opérationnelles que le Sénat formule ?

de reconnaissance (PFR) versée aux sapeurs-pompiers volontaires a fait économiser 30 millions d'euros à l'État. Il était convenu que cet argent soit reversé aux SDIS pour investir dans le domaine de la sécurité des pompiers.

Les Républicains. CETA vous, monsieur le Premier ministre, que j'adresse cette question. CETA, quatre lettres qui résonnent comme une question controversée dans la tête des Français. CETA l'Assemblée nationale que le texte a été ratifié en juillet, malgré la bronca qu'il a suscitée, y compris au sein de votre propre majorité. CETA quelle date, monsieur le Premier ministre, que vous allez enfin programmer l'étude du texte de ratification devant le Sénat ?

que vous allez continuer d'ouvrir les portes, créant une concurrence déloyale pour nos produits. C'est de tout cela que les Français ne veulent plus ! Alors, CETA vous, monsieur le ministre, que je demande de prendre vos responsabilités dans cet hémicycle, devant les représentants des Français. Annoncez vite la date exacte de l'examen au Sénat du CETA ! Cela vous honorerait

Depuis mon arrivée au Sénat en 2014, je n'ai eu de cesse d'alerter les gouvernements successifs sur la situation du centre hospitalier Louis-Constant-Fleming de Saint-Martin. Mes interpellations portaient soit sur la situation financière et budgétaire, soit sur les conditions d'exercice de la médecine et la qualité des soins. Madame la ministre, je vous ai régulièrement tenue informée, au travers de questions d'actualité au Gouvernement ou par courrier, de situations qui ne peuvent me laisser insensible. Je tiens d'ailleurs à vous renouveler mes remerciements pour les réponses apportées aux difficultés apportées aux difficultés des médecins urgentistes. Récemment, un infirmier-anesthésiste a tenté de mettre fin à ses jours au sein même du bloc opératoire. Ce nouveau drame illustre, une fois encore, la tension exacerbée qui règne au sein du personnel médical du centre hospitalier. (ARS) a été sensibilisée ; un changement de direction a été effectué et une administration provisoire a été mise en place. Pour autant, force est de constater que la situation est devenue insoutenable. Aussi, madame la ministre, avec toutes les réserves et précautions d'usage, pouvez-vous rassurer la population saint-martinoise ? Que comptez-vous faire pour que la qualité des soins et la sécurité des patients soient garanties,

Je comprends l'inquiétude dont vous vous faites le porte-parole aujourd'hui. Le drame dont vous vous faites l'écho ne peut que nous alerter et nous émouvoir. Deux ans après le passage de l'ouragan Irma sur votre île, la reconstruction est toujours en cours, à l'hôpital comme pour d'autres structures. Vous l'avez rappelé, le centre hospitalier Louis-Constant-Fleming a été placé sous administration provisoire depuis le mois d'avril dernier. Cette décision a été prise face à la situation extrêmement dégradée de l'établissement en matière de trésorerie et de recouvrements. Il y avait aussi des conflits récurrents en interne. Mes services ont pu prendre connaissance des premières conclusions de l'administration provisoire voilà quelques semaines. Un certain nombre de dysfonctionnements ont été identifiés et confirmés. Il nous faut maintenant apporter des solutions. Je pense, par exemple, à la rédaction d'un projet médical, qui n'existe pas pour l'île de Saint-Martin. Le centre hospitalier dispose d'atouts très importants en matière de compétences médicales et chirurgicales. J'avais eu l'occasion de rencontrer les personnels dans la semaine qui a suivi Irma, et j'ai pu me rendre compte de leur engagement, alors qu'il y avait des pillages et que l'hôpital était Je le rappelle, il s'agit du principal établissement sur l'île. Je sais qu'un grand nombre de professionnels de cet établissement y sont attachés et qu'ils sont capables de faire des efforts afin d'assurer sa pérennité.

de l'administration provisoire. Vous pouvez compter sur ma vigilance. Il est primordial que les Saint-Martinois retrouvent la confiance dont ils ont besoin.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, il y a un décalage permanent entre le discours, recouvert d'un vernis social, du Gouvernement, et la réalité, qui n'est que celle d'un triste libéralisme à tous crins. Ces derniers jours, voire ces dernières heures, des millions de Français ont compris que le vrai sens des initiales LREM, c'était « La Retraite En Moins » ... probablement pour privatiser plus Au début du quinquennat, on aurait pu parier sur de la maladresse, comme pour les 5 euros pris au titulaire de l'APL, alors que les Français les plus riches gagnaient chacun 1,7 million d'euros par an avec la Quant à la suppression de la taxe d'habitation, c'est 8 milliards d'euros pour les 20 % les plus aisés et 0 euro pour les 20 % les plus pauvres. Cette mesure, présentée comme sociale, fragilisera avant tout les collectivités. que dire de la désindexation des prestations sociales ou de la réforme de l'assurance chômage, qui fera 1,3 million de perdants ? Il semble donc qu'avec vous, socialement, il y a toujours des vaincus et des vainqueurs, mais vous n'êtes au chevet que des derniers. Avec vous, l'État est comme amputé de sa main gauche, celle de l'État-providence. Je souhaite aborder un exemple révélateur, en caressant l'espoir que vous me démentirez. Lors des assises de l'eau de 2018, le Premier ministre a annoncé la volonté de l'exécutif « d'accélérer le déploiement de la tarification sociale de l'eau à destination des populations les plus fragiles » et la mise en place d'un chèque eau, sur le modèle du chèque énergie. Là encore, beau discours, utile, d'autant que le nombre de Français pour lesquels la facture d'eau et d'assainissement dépasserait le seuil d'acceptabilité est estimé à 2 millions. La généralisation de la tarification sociale de l'eau a été adoptée au Sénat et à l'Assemblée nationale, mais le chèque eau s'est, si j'ose dire, évaporé du dispositif, et la loi de finances n'a pas corrigé cet oubli. cet oubli. Madame la secrétaire d'État, comment allez-vous accompagner les collectivités locales dans la généralisation de la tarification sociale de l'eau pour lutter contre la précarité hydrique ? Allez-vous mettre en place un chèque eau ou faire supporter aux collectivités locales vos ambitions sociales, bref, faire payer la solidarité par les autres ?

par an et par ménage, et beaucoup de dispositions diverses- chèques, remises, accompagnements particuliers pour les économies d'eau -développées par les collectivités territoriales.

à l'unanimité, et la commission mixte paritaire se réunit précisément aujourd'hui à dix-sept heures. J'espère que cette disposition sera maintenue. La tarification sociale de l'eau d'un service public assuré par les collectivités territoriales, comme vous le savez, et vous êtes, comme nous, attachés à la libre administration des collectivités locales. Autant nous pouvons aider chaque collectivité à trouver ses modalités de généralisation,

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la ministre du travail, à laquelle je souhaite un prompt rétablissement. Madame la ministre, votre gouvernement a décidé de reprendre la main sur le pilotage de l'apprentissage au niveau national en supprimant toute régulation, fonction qui était exercée par les régions. Aujourd'hui, l'Association des régions de France (ARF) tire la sonnette d'alarme sur l'évolution des choix d'orientation sur les métiers, qui tend à accentuer l'inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Cela ne va pas contribuer à régler le problème crucial des postes non pourvus. Madame la ministre, allez-vous prendre cette situation en compte et redonner un pouvoir de régulation aux régions, qui, en raison de leur compétence économique, pourraient travailler avec les branches professionnelles et anticiper en orientant les choix de formation sur les métiers créateurs d'emplois ? Aujourd'hui, la réalité, c'est que les entreprises peinent à recruter. Les candidats à l'apprentissage se retrouvent devant de multiples interlocuteurs et ont du mal à entrer dans les dispositifs. Les apprentis les plus défavorisés ont besoin d'un accompagnement pour trouver un employeur, trouver un hébergement et faire les démarches afin d'obtenir les aides nécessaires. Pour finir, où en êtes-vous des négociations qui doivent s'engager avec les régions de France sur les compensations que, d'après leurs comptes, vous leur devez ?

de colère que je me permets de rectifier ou de compléter vos informations. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, promulguée le 5 septembre 2018, est déjà largement en vigueur, et produit de premiers résultats. Nous sommes d'accord, il ne s'agit que des premiers résultats,

Toutes les simplifications pour les entreprises- l'aide unique, l'embauche tout au long de l'année, les horaires de travail, les conditions de travail -sont en vigueur depuis le 1 janvier, ainsi que toutes les aides aux apprentis, permis

puisque plus de 500 CFA se sont enregistrés depuis le début de l'année. De la même façon, le coût au contrat est déjà en application. Il a été avancé de trois mois, car les CFA nous l'ont demandé. Les entreprises, les jeunes et les CFA plébiscitent cette réforme. de 27 % du nombre d'apprentis chez les compagnons, de 17 % dans les maisons familiales rurales, de 10 % dans l'industrie. Nous avons un seul sujet : les 500 millions d'euros que le Premier ministre s'est engagé à transférer aux régions le seront dès que l'Association des régions de France aura proposé cette répartition. OEuvrons ensemble

Madame la ministre, comme le Sénat vous l'avait proposé lors de nos débats sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, je vous demande solennellement de revoir votre position et de redonner aux régions une vraie compétence de régulation. Vous demandez aux régions de s'investir et, en même temps, vous leur retirez une compétence. C'est d'une incohérence totale ! Il faut absolument que cette compétence de régulation et d'accompagnement revienne aux régions. En raison de leur compétence économique, et dans l'esprit d'une nouvelle étape de la décentralisation,

La séance est reprise. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote, présentée par Mme Valérie Létard et plusieurs de ses collègues (proposition n°

alertée par des élus locaux du Nord de l'explosion du phénomène de consommation détournée du protoxyde d'azote chez les jeunes, j'ai pu constater l'ampleur de la consommation de ce gaz hilarant dans l'espace public et l'importance de la diffusion de ce À l'évocation d'un « gaz hilarant », on pourrait imaginer un sujet léger, mais il n'en est rien ! L'usage par inhalation du protoxyde d'azote, connu depuis longtemps, est en augmentation significative chez les jeunes. Utilisé dans le champ médical pour ses propriétés anesthésiques et analgésiques, le protoxyde d'azote est aussi employé comme gaz de pressurisation pour les siphons à crème chantilly. Le protoxyde d'azote fait malheureusement aussi l'objet d'usages détournés en raison de son effet euphorisant. devenu le troisième produit psychoactif le plus consommé chez les jeunes. Son inhalation s'est largement banalisée et devient pour de nombreux jeunes, notamment mineurs, une première expérience de consommation addictive, avec- on ne le sait que trop peu -des conséquences désastreuses pour la santé, selon les quantités et la fréquence de sa consommation. Voilà un an, le rapport de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies relevait une évolution de l'usage et de la consommation du protoxyde d'azote, avec son irruption dans l'espace public. Alors qu'il était réservé jusqu'alors aux milieux festifs alternatifs, tels que les teknivals, nous assistons depuis deux ans à une banalisation de la consommation de ce produit : de nombreuses petites cartouches grises contenant le gaz sont retrouvées, de façon continuelle et en quantité importante, dans l'espace public de nombreux territoires.

Nouvelle drogue à la mode, ce gaz fait fureur chez les jeunes majeurs, mais aussi chez les mineurs adolescents- collégiens comme lycéens -, et on constate une véritable addiction à son effet euphorisant. Accessible librement pour son usage domestique, il est vendu dans les commerces de proximité, épiceries, supermarchés, certains bars qui mettent en avant ces cartouches comme des produits d'appel ou sur internet, sans aucune restriction, et à un coût relativement modique- entre 30 centimes et 1 euro la cartouche. On en trouve aussi dans les établissements de type discothèques, bars de nuit, qui vendent à côté des alcools, des ballons de protoxyde à des prix constatés entre 3 et 5 euros le ballon. En l'état actuel de notre droit, nous sommes donc face à un phénomène de consommation d'ampleur d'un produit psychoactif, loin d'être anodin, et face à un phénomène d'addiction facilité par une commercialisation ordinaire du produit, sans pouvoir ni agir, ni protéger les mineurs de ces comportements à risques, ni prévenir les problèmes sanitaires. Cela nous renseigne sur plusieurs points. Tout d'abord, le caractère récréatif du produit le consacre auprès des consommateurs jeunes comme un produit non dangereux, ce que renforce l'absence de visuel ou de pictogramme sur l'emballage, que cela permettrait de caractériser sa dangerosité. Ensuite, la banalisation même de ce produit auprès d'un public jeune est en cours, puisqu'aujourd'hui des cartouches sont retrouvées aux abords des collèges et lycées et qu'un business avec commerce de revente s'organise parfois.

Par souci de clarté du message juridique, nous avons estimé qu'il fallait que la prévention puisse se faire autant en amont, c'est-à-dire au stade de la vente, qu'en aval. Il nous a semblé important que l'incitation à la consommation soit considérée comme répréhensible, pour répondre au contournement de l'acte d'achat, au business de la revente ou encore au marché qui se développe, associant ballons de baudruche et contenants plus importants de protoxyde d'azote. Pour rendre opérant ce texte, la commission a maintenu le principe de ce double filtre en proposant d'utiles aménagements. Par ailleurs, nous avons estimé que, pour contrer l'image festive du protoxyde d'azote, la réglementation en matière d'affichage sur le contenant devait évoluer et que la prévention devait être auprès des populations jeunes pour leur exposer les conséquences sanitaires de l'inhalation de ces produits. Je retrouve avec le texte de la commission l'esprit qui était le nôtre lors de l'écriture de la proposition de loi.

légiférer, parce que c'est devenu un problème de santé publique. Les médecins sont clairs sur ce point : les dangers de l'inhalation du protoxyde d'azote sont bien réels, qu'ils soient immédiats ou à plus long terme en cas d'utilisation régulière. Le protoxyde d'azote n'étant pas métabolisé par l'organisme, ses utilisateurs se sentent souvent parfaitement normaux dans les deux minutes suivant l'inhalation, ce qui les conduit à poursuivre leur consommation. La dimension addictive du protoxyde d'azote dans son usage détourné ne fait aucun doute. De plus, brûlures par le froid du gaz libéré, détresse respiratoire, asphyxie, vertiges, maux de tête, vision floue, malaises, crise de panique, problèmes cardiaques peuvent survenir. En outre, la consommation excessive de ce produit a des effets graves sur la santé, qu'ils soient psychiques, neurologiques ou encore liés à un déficit en vitamine B12, à l'origine d'une sclérose de la moelle épinière pouvant être irréversible.

avec l'Union européenne afin d'affiner la rédaction juridique des dispositions qui permettront de faire évoluer la réglementation, considérant le protoxyde d'azote comme un produit dangereux, comme c'est le cas pour son usage médical.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comme beaucoup de nos concitoyens, c'est grâce à Valérie Létard et à ses collègues que j'ai découvert- avec un certain étonnement, je dois le dire -la dernière pratique psychoactive à la mode chez les jeunes Français inhaler le gaz contenu dans les petites cartouches destinées aux siphons à crème chantilly pour en obtenir, pendant quelques minutes à peine, des effets semblables à l'ivresse. Passé l'étonnement, je me suis rappelé que les Français avaient détenu pendant quelques années le record de la consommation d'antidépresseurs en Europe et qu'ils restaient champions de la consommation de cannabis. Ce n'est sans doute pas le moment d'examiner ce que de telles pratiques disent de l'état psychologique d'une population ou de spéculer sur l'avenir qu'elles promettent à sa jeunesse, mais j'invite chacun ici à accorder à ces questions ne serait-ce qu'un instant de réflexion, avant que nous envisagions de blâmer, de prévenir, d'empêcher ou de punir. Souvenons-nous simplement que les usages de substances psychoactives font partie des expérimentations auxquelles se livrent tous les adultes en devenir, à toutes les époques, et sont à replacer dans un contexte et une histoire. du protoxyde d'azote est d'ailleurs assez intéressante. En effet, l'usage qu'en font les jeunes d'aujourd'hui est vieux de deux siècles. Les propriétés médicales et euphorisantes du protoxyde d'azote sont établies à la fin du XVIII siècle par un chimiste anglais. C'est ce même scientifique qui organisa les premiers usages récréatifs collectifs de ce gaz, à l'été de 1799, et en devint lui-même dépendant. L'engouement pour le protoxyde d'azote ne s'est pas démenti jusqu'à la fin du XIX siècle. On peut faire l'hypothèse qu'ensuite c'est la concurrence d'autres substances qui l'a fait passer au second plan et lui a laissé l'image d'un produit relativement anodin. Alors que ce produit n'était plus utilisé qu'en médecine et dans des conditions très encadrées, son usage récréatif fait l'objet d'un emballement nouveau depuis la fin des années 1990 dans les milieux festifs alternatifs et, depuis le milieu des années 2010, chez les jeunes de tous les milieux. Songez qu'à présent les collégiens s'en voient proposer à la sortie de leur établissement scolaire. d'azote peut s'expliquer assez facilement. D'abord, le protoxyde d'azote est légal et, par conséquent, très facile d'accès. Vendu généralement dans de petites cartouches d'aluminium conditionnées par boîtes de cinq, dix ou vingt destinées à faire fonctionner les siphons à usage culinaire culinaire dont ont besoin les amateurs d'émulsions de toutes sortes, ce gaz se trouve au rayon cuisine de tous les commerces. Son mode d'administration est simple : le gaz est transféré dans un ballon de baudruche, puis inhalé au rythme de la respiration. Ensuite, ce produit est très peu onéreux. Rendues omniprésentes par la mode télévisuelle de la cuisine créative, les cartouches coûtent environ 1 euro pièce, souvent moins. Surtout, la hausse de la demande a attiré sur le marché de nouveaux entrants, qui vont jusqu'à proposer sur internet des bonbonnes entières à prix cassé et dont la réclame annonce fièrement que les ballons de baudruche sont offerts avec la livraison- ne laissant aucun doute sur l'usage qui sera fait du produit. En outre, les effets du protoxyde d'azote sont brefs, de l'ordre de quelques minutes seulement, et difficiles à détecter. Il est par conséquent plus commode, avant de se rendre en classe ou de rentrer dîner chez ses parents, d'inhaler du protoxyde d'azote que de fumer du cannabis, si l'on souhaite éviter d'attirer l'attention. Enfin, la popularité du protoxyde d'azote s'explique assez largement par le fait qu'il s'agit d'une mode, venue des pays anglo-saxons, via les Pays-Bas et la Belgique, mais aussi propagée par les réseaux sociaux. C'est toutefois très abusivement que l'on parle de « gaz hilarant », car les effets du protoxyde d'azote sur la santé n'ont pas de quoi faire rire. Sa manipulation elle-même est dangereuse, car c'est un gaz froid, qui peut occasionner des brûlures. Même inhalé avec précaution, il produit des effets qui ne sont pas sans danger pour les consommateurs et leur entourage : distorsion visuelle

Surtout, en consommation chronique, le protoxyde d'azote interfère dans le métabolisme de la vitamine B12, indispensable au bon entretien de la gaine de myéline qui protège les nerfs. En d'autres termes, les consommateurs de grandes quantités de protoxyde d'azote risquent des atteintes extrêmement graves de la moelle épinière.

leur consommation s'élevait à plusieurs centaines de cartouches par jour pendant un à trois mois. Cinq cas sont en outre en cours d'examen pour des symptômes analogues ; ceux dont l'âge nous a été communiqué ont respectivement 23, 19, 18 et 17 ans. ans. Que faire ? Laisser passer la mode ? Faire confiance aux parents ? Se contenter de communiquer sur la dangerosité du produit ? Le Gouvernement semble avoir fait ce dernier choix, en publiant un communiqué le 19 novembre dernier. Pour l'heure, les maires de nos communes sont seuls en première ligne pour tenter de juguler le phénomène. Des arrêtés interdisant la vente ou l'usage de protoxyde d'azote à des fins récréatives ont été pris dans pas moins de 47 communes, du Nord à l'Hérault, en passant par la Seine-Saint-Denis. Outre les problèmes de santé publique, l'usage détourné de ce gaz cause de réels troubles à l'ordre public. La seule commune de Loos, où je me suis rendue et qui compte 21 000 habitants, envoie chaque mois au recyclage 100 kilogrammes de cartouches d'aluminium retrouvées sur la chaussée ! Depuis peu, les jeunes sont passés à la vitesse supérieure, puisque l'on retrouve aussi des bonbonnes dans les lieux publics. Les arrêtés ont leurs limites. Ils sont territorialisés, donc contournables, ou impraticables dans les grandes agglomérations. Ils varient selon les communes et ils sont parfois fragiles juridiquement. Observons par ailleurs qu'un nombre croissant de pays confrontés avant nous à ce phénomène ont fait le choix de légiférer pour interdire la vente aux mineurs, voire la simple possession de protoxyde d'azote à des fins récréatives de plus en plus d'États américains, d'États australiens, le Royaume-Uni, Chypre, la Croatie ou encore la Corée du Sud. Avant-hier encore, les Pays-Bas, qui avaient jusqu'à présent tout misé sur la prévention, ont annoncé s'engager dans cette voie. Enfin, j'avoue craindre que le phénomène ne se répande, comme beaucoup de modes importées des pays anglo-saxons. Je fais d'ailleurs observer qu'au Royaume-Uni, depuis 2001, on recense 36 jeunes personnes mortes Cette proposition de loi, cosignée par plus de quatre-vingt-dix de nos collègues siégeant dans toutes les travées, fait donc, après de nombreux autres pays, trois choses assez simples. D'abord, elle interdit la vente aux mineurs du protoxyde d'azote, en commerces physiques comme dans les lieux publics ou en ligne. Ensuite, elle pénalise la provocation d'un mineur à la consommation de ce type de substance. elle entend contribuer à la prévention, en obligeant les fabricants à faire apparaître la dangerosité du gaz sur les contenants et en renforçant l'information sur internet et à l'école- grâce aux amendements de M. Grand. On nous objectera peut-être que ce texte pénalise une filière. Il faut savoir que les industriels que j'ai auditionnés soutiennent cette initiative. On nous objectera éventuellement qu'il faudrait interdire le protoxyde d'azote tout court. Cela s'entend, mais c'est une substance pour l'heure irremplaçable en cuisine et, s'il fallait interdire chaque objet dont le mésusage peut provoquer des catastrophes, nous n'aurions hélas ! pas fini de siéger. On nous objectera sans doute que la mode du protoxyde d'azote sera chassée par une autre, qui appellera un texte à son tour, et qu'il est vain de légiférer par saccades. C'est très juste. La commission des affaires sociales a donc ouvert un nouveau livre dans le code de la santé publique consacré aux usages détournés dangereux de produits de consommation courante. Très bien ! Elle a également élargi le délit prévu à l'article 2 à toute provocation d'un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante courante pour en obtenir des effets psychoactifs. Pourraient ainsi être couvertes, à l'avenir, d'autres substances, tel l'hélium qui, au Royaume-Uni, tue quatorze fois plus encore que le protoxyde d'azote. On nous objectera encore que cette proposition de loi vise à protéger les mineurs, alors que les cas sanitaires les plus graves sont observés chez de jeunes majeurs. C'est encore vrai, mais c'est attribuer à cet humble texte les objectifs de la politique de santé publique tout entière. Le législateur n'a pas le pouvoir d'empêcher quiconque de faire un usage autodestructeur d'un produit de consommation courante. Qui comprendrait, en revanche, qu'il ne cherche pas à retarder le contact des mineurs avec une substance dont l'usage détourné est notoirement addictif et nocif ? On nous objectera enfin que l'interdiction de vente aux mineurs est difficile à faire respecter. C'est toujours vrai, mais que ferait-on s'il fallait systématiquement conclure de la difficulté à l'impossibilité ? Qui souhaiterait ici revenir sur l'interdiction de vente de tabac et d'alcool aux mineurs, au seul motif que son application est périlleuse ? En réfutant ces objections, je ne prétends nullement que cette proposition de loi soit parfaite. J'entends simplement pointer du doigt les limites de notre pouvoir de législateur, tant que le protoxyde d'azote restera considéré comme un produit d'usage courant. Il y a en effet quelque paradoxe à observer que la version médicale de cette substance, le Méopa, est considérée comme un stupéfiant alors qu'elle est mélangée à parité avec de l'oxygène et utilisée de manière très encadrée, tandis que sa version pure est accessible aux enfants. Sans doute M. le secrétaire d'État nous précisera-t-il ce que le Gouvernement compte faire en urgence pour mieux encadrer ce produit, dont l'usage culinaire, qui justifie sa commercialisation large, est de longtemps postérieur à son usage récréatif, même si celui-ci est resté mal connu en dehors de son pays de naissance, le En attendant qu'un changement de classification réglementaire du protoxyde d'azote aboutisse, nous serions infiniment heureux que le Gouvernement contribue à améliorer ce texte et qu'il s'engage formellement devant nous à ce que la navette parlementaire puisse aller à son terme dans les délais les meilleurs et les plus compatibles avec nos obligations européennes. Mes chers collègues, il était devenu urgent d'agir, comme élus locaux, comme parents et comme législateurs, pour endiguer la multiplication de ces comportements à risque. La parole

vise à protéger les mineurs contre les usages dangereux du protoxyde d'azote. Vous le savez, la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, est pleinement engagée dans la prévention des consommations à risque et dans la lutte contre les addictions, engagement que je partage pleinement, en particulier pour protéger les plus jeunes. Avec le plan Priorité prévention lancé en mars 2018 et ses deux plans thématiques de lutte contre le tabac et de mobilisation contre les addictions, nous avons fixé un cap ambitieux afin de lutter contre les consommations à risque,

de façon discontinue des usages détournés de protoxyde d'azote en milieu festif. Si la consommation de protoxyde d'azote ne fait pas l'objet d'un suivi en tant que tel en population générale adulte et adolescente, elle est bien prise en compte au titre des données de consommations. En 2017,

Ces éléments suffisent à considérer qu'il s'agit d'un problème sanitaire devant faire l'objet de mesures de protection. Aussi le Gouvernement partage-t-il les objectifs de ce texte, qui sont de protéger les jeunes consommateurs de protoxyde d'azote

pour le travail réalisé depuis. Dès le mois de mai, le Gouvernement a informé les préfectures et incité les acteurs régionaux à se rencontrer pour échanger sur les actions pouvant être mises en oeuvre sur le territoire. Il y a quelques semaines, le ministère des solidarités et de la santé a diffusé un message auprès du grand public pour l'informer sur le phénomène, sur les actions mises en place et sur celles qu'étudient les autorités sanitaires. En parallèle, les dix-sept agences régionales de santé santé ont reçu les éléments d'information et de gestion leur permettant de mettre en place des actions de prévention, de favoriser le diagnostic et la mise en place d'une prise en charge thérapeutique rapide et adaptée des usagers concernés, de renforcer le signalement des cas et la diffusion de messages de vigilance aux usagers. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette proposition de loi, dont l'objectif de protection des plus jeunes est évidemment tout à fait légitime. Nous devons être lucides : l'interdiction de la vente aux mineurs ne permettra pas, à elle seule, à elle seule, de mettre fin aux pratiques de détournement d'usage de produits de consommation courante et de protéger nos jeunes. Les difficultés de respect de l'interdiction de la vente des produits du tabac et de l'alcool aux mineurs,

De plus, et il est important de le souligner, les intoxications graves observées en France, vous l'avez dit, madame la rapporteure, concernent principalement de jeunes adultes. La mesure aurait donc peu d'effets sur ce public. Il nous faut aussi réfléchir à ce qui peut être fait pour le public des jeunes majeurs. La proposition de loi initiale prévoyait l'apposition d'un pictogramme sur les cartouches de protoxyde d'azote rappelant l'interdiction de vente aux mineurs, auquel vous avez substitué en commission une mention indiquant la dangerosité du produit à apposer sur les conditionnements. Cette mention nous semble en effet plus appropriée pour signaler le danger lié à l'inhalation du protoxyde d'azote et répondre à l'objectif d'information de tous sur les risques associés à des usages détournés du produit. Par ailleurs, à la différence de la consommation du tabac et de l'alcool chez les jeunes, le protoxyde d'azote soulève la question plus générale de l'appréhension et de l'encadrement de l'usage détourné de produits de consommation courante

produits. En commission, vous avez élargi l'infraction d'incitation aux usages détournés dangereux de produits de consommation courante. C'est une bonne chose, même s'il nous faudra sûrement encore poursuivre la réflexion pour sécuriser cette disposition. Nous aurons l'occasion d'y revenir à l'occasion de l'examen de votre amendement,

À côté de ces mesures normatives, nous devons continuer à travailler, aussi et sans doute surtout, madame la rapporteure, sur la prévention des usages détournés, par une meilleure information des jeunes sur les risques associés, dans une approche globale de prévention des consommations de tous les produits psychoactifs.

Nous devons donc informer sur les risques réels des usages détournés en général et de la consommation de substances psychoactives et ne pas uniquement focaliser nos messages sur le seul protoxyde d'azote. Ces actions passent en priorité par l'école, l'école, par les universités- je l'ai dit, les jeunes majeurs sont des consommateurs -, par les acteurs proches des jeunes. La modification du code de l'éducation que vous avez effectuée en commission va dans ce sens. Il nous faut aussi également mieux faire connaître les dispositifs d'aide mis à disposition des jeunes, de leur entourage et du public en général, pour toutes les questions ou difficultés liées à la consommation de produits ou de drogues. C'est aussi l'objet du plan Priorité prévention que j'ai évoqué au début de mon intervention. Je pense en particulier aux Consultations jeunes consommateurs,

et d'échanges. Mesdames, messieurs les sénateurs, notre souhait commun est bien d'agir face à l'importance de cette problématique sanitaire, sur laquelle les leviers d'action sont complexes et multiples. Nous saluons l'initiative de cette proposition, et nous souhaitons poursuivre le travail pour parfaire collectivement le dispositif proposé.

du protoxyde d'azote. Je salue l'initiative de notre collègue Valérie Létard, dont je partage pleinement les objectifs. Depuis janvier 2019, dix cas graves, dont huit dans les Hauts-de-France, ont été recensés, suite à l'inhalation de cette substance par des mineurs. Le protoxyde d'azote, aussi connu sous le terme de « gaz hilarant », est sans doute l'agent volatile le plus ancien de la pharmacopée anesthésique. Ses propriétés euphorisantes, découvertes en 1799 par le chimiste anglais Humphry Davy, ont par la suite largement contribué au progrès de l'odontologie et de la chirurgie. Si ce produit est encore utilisé en chirurgie, en complément de produits anesthésiants, il est également employé en tant que gaz de pressurisation en cuisine, dans les siphons pour crème chantilly. De même, son usage reste récurrent dans le monde sportif, afin de soulager les douleurs et les blessures des athlètes durant leurs performances. Ce produit peut être acheté, pour une somme modique, par n'importe qui, en supermarché ou sur internet. Sa facilité d'accès et la publicité sur ses effets hilarants diffusée sur les réseaux sociaux ont popularisé un usage détourné, comme s'il s'agissait d'un produit purement récréatif et festif, chez des mineurs de plus en plus jeunes. Sa consommation, souvent en groupe, peut atteindre jusqu'à 200 capsules par jour. Le gaz a une action immédiate et agit sur une courte durée, provoquant des crises de fou rire et des modifications des perceptions.

Sa consommation chronique provoque des carences en vitamine B12 susceptibles d'entraîner des dommages irréversibles sur le système nerveux central et la moelle épinière. Cela a été rappelé, notamment par Valérie Létard. De nombreuses études scientifiques à travers le monde convergent sur les conséquences neurologiques de l'inhalation sans contrôle sans contrôle de trop fortes doses. La Grande-Bretagne recense huit décès par an directement liés à la consommation de cette drogue. Le problème arrive en France, en particulier dans la métropole lilloise. Aussi, à la fin du mois de septembre, le maire de Tourcoing a pris un arrêté municipal pour en interdire l'usage détourné chez les mineurs. Les villes de Roncq et Neuville-en-Ferrain ont suivi, alertées par les familles et les nombreuses capsules vides jonchant les trottoirs. Il semblerait que certains commerçants vendent directement les capsules contenant cette substance avec les ballons de baudruche qui servent à leur inhalation.

Pour accompagner cette mesure, des campagnes d'information sur les risques de cet usage détourné sont prévues dans les établissements scolaires. Quant aux industriels, ils seront tenus d'apposer sur chaque contenant incluant ce produit un pictogramme indiquant l'interdiction de vente aux moins de 18 ans. 18 ans. Toutes les actions de sensibilisation auprès des mineurs, y compris par des personnes célèbres, sont une bonne chose. Nous soutenons l'ensemble de ces dispositions, qui vont permettre de protéger les mineurs, vulnérables et influençables, des risques liés à l'inhalation de protoxyde d'azote en limitant sa banalisation en France.

la proposition de loi déposée au mois d'avril 2019 par Mme Valérie Létard et quatre-vingt-quatorze de nos collègues tend à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote.

en lien avec l'usage détourné du protoxyde d'azote. Cette annonce suivait de près le communiqué de l'Association française des centres d'addictovigilance du 5 novembre intitulé.

Or nous ne pouvons qu'être surpris par l'extrême facilité avec laquelle il est possible de s'en procurer. Je souhaite alerter et insister sur ce point

La question se pose de la responsabilité des fabricants et des revendeurs, qui pourraient être considérés comme complices de l'usage détourné du protoxyde d'azote.

Ces sites devraient également être contraints de signaler les nombreux dangers d'une utilisation non conforme : dépendance, risques psychiques, neurologiques et cardio-vasculaires. La liste est longue, des nausées et vomissements à l'asphyxie, des troubles hématologiques sévères à l'addiction. Si le phénomène touche le plus dramatiquement le département du Nord et les Hauts-de-France, la jeunesse de la région Occitanie est également très concernée.

qui a bien saisi les enjeux de santé publique et les risques sanitaires. Elle mène des actions de prévention, d'alerte et de vigilance, notamment à destination des parents. Les deux phénomènes vraiment nouveaux sont la jeunesse toujours plus grande des consommateurs, ainsi que la répétitivité de l'usage et sa chronicisation, avec tous les risques induits inacceptables. Il faut cesser de placer ce gaz

S'il devient nécessaire de légiférer, de poser un cadre pour limiter les dérives, c'est bien parce que la consommation récréative de protoxyde d'azote, détournée donc de ses usages originels, est une pratique qui se répand, particulièrement dans le Nord de la France. Utilisé dans le domaine médical pour pratiquer des anesthésies et dans la vie courante, notamment dans les siphons servant à faire de la crème chantilly, ce gaz, par les sensations euphorisantes qu'il procure, séduit de plus en plus d'adeptes, principalement des jeunes. Comme en témoigne son surnom de gaz « hilarant », ce produit jouit d'une image positive. Légal, il ne fait actuellement l'objet d'aucune restriction à la vente. Il est facilement disponible sur internet, mais aussi dans les commerces de proximité, les supermarchés. Il est très bon marché et coûte moins de 1 euro la cartouche. D'où sa triste popularité ... Une étude de la mutuelle étudiante Smerep, dévoilée l'an dernier, classait le protoxyde d'azote au troisième rang des drogues les plus consommées par les étudiants, derrière le cannabis et le poppers. Drogue tendance, ce gaz fait donc fureur chez nos jeunes, créant une véritable dépendance à l'effet euphorisant. Aucun visuel ou pictogramme sur l'emballage n'alerte sur les dangers d'inhalation de ce produit. Pourtant, comme le souligne plusieurs études scientifiques, et comme le rappelait il y a moins d'un mois les autorités sanitaires, l'usage détourné du protoxyde d'azote expose à des risques majeurs. des risques immédiats tout d'abord : asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlures par le froid du gaz expulsé de la cartouche, notamment. Plus grave encore, lorsqu'il est consommé de manière régulière et/ou à forte dose, les médecins parlent de carence en vitamine B12, d'anémie, d'atteinte de la moelle épinière et de toxicité directe sur les cellules nerveuses pouvant entraîner des dégâts neurologiques définitifs. La consommation associée à d'autres produits, comme l'alcool, majore bien évidemment ces risques. Depuis le début de l'année, vingt-cinq signalements d'effets sanitaires sévères ont été enregistrés en France, dont dix cas graves avec des séquelles pour certains, comme des paralysies des membres, à des degrés divers. En Grande-Bretagne ou aux États-Unis, où le phénomène est plus ancien, le protoxyde d'azote tue. On comprend mieux pourquoi de plus en plus d'États dans le monde restreignent la vente et l'usage récréatif de ce gaz. Si, dans son usage détourné, ce gaz provoque en quelques inspirations un fou rire irrépressible, on voit bien qu'il devient urgent de débanaliser une pratique, qui n'a décidément rien d'hilarante, et de faire des propositions, sans pour autant mettre en oeuvre une politique de répression ou d'interdiction d'un produit domestique et médical, dont l'usage reste indispensable. Aujourd'hui, comme trop souvent, les maires se retrouvent seuls, en première ligne, pour faire face à ce phénomène. Ils sont contraints de prendre des arrêtés pour interdire la vente aux mineurs ou la consommation de protoxyde d'azote afin de faire cesser des troubles à la sécurité, à la tranquillité ou à la salubrité publiques. à la salubrité publiques. Les limites de tels arrêtés sont évidentes : ils ne peuvent s'appliquer que s'il existe une force publique pour constater les infractions. En outre, rien n'empêche évidemment les consommateurs d'aller acheter des cartouches dans les communes voisines. alors secrétaire d'État à la santé, envisageait déjà de restreindre la vente de protoxyde d'azote aux seuls utilisateurs industriels. La législation n'a malheureusement pas évolué depuis. La mesure phare du texte examiné ce jour est l'interdiction de vendre ce gaz aux mineurs, y compris sur les sites de commerce en ligne. Les industriels auraient en outre l'obligation de mentionner sur l'emballage la dangerosité du protoxyde d'azote. Il est également prévu de pénaliser le fait d'inciter un mineur à faire un usage détourné de ce produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs. vont dans le bon sens, comme tout ce qui permettra de renforcer la prévention en direction de nos jeunes, collégiens et lycéens, notamment. Pour les sénateurs du groupe socialiste et républicain, dont certains sont aussi des parents, des élus locaux, cet encadrement législatif va dans le bon sens. C'est pourquoi, vous l'aurez compris, mes chers collègues,

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, nous voici réunis pour évoquer et tenter de contenir une pratique qui s'étend chez les jeunes Français de tous les milieux, alors qu'elle sévit et fait des ravages depuis de nombreuses années, voire des décennies, dans d'autres pays. Le protoxyde d'azote, connu depuis les années 1800, est utilisé en cuisine dans les siphons et en médecine pour ses propriétés anesthésiques et analgésiques. Jusque-là, il n'y a rien à reprocher à ce gaz, qui remplit parfaitement ces deux fonctions. Malheureusement, certaines personnes en recherche de sensations fortes l'ont détourné de son usage traditionnel pour en obtenir des effets psychoactifs, que l'on peut comparer à ceux des drogues ou de l'alcool. Ce détournement pose plusieurs problèmes, qui appellent la mobilisation des pouvoirs publics et justifient la discussion de ce jour.

où onze personnes, peut-être plus, ont déjà déclaré des troubles neurologiques graves dus à ce gaz. Face à cela, les municipalités ne peuvent que prendre des arrêtés qui ne résolvent rien. L'incapacité des pouvoirs publics à lutter contre cette consommation croissante est notamment liée à la facilité d'accès des jeunes au protoxyde d'azote. Cela a été rappelé : n'importe qui peut en acheter à moindre coût dans le commerce, sous la forme de cartouches destinées aux siphons. Sa consommation est rapide et ne laisse aucune trace, contrairement aux joints dont l'odeur peut alerter les parents ... Ce qui explique Ce qui explique surtout le succès de ce gaz, c'est la méconnaissance totale qui perdure sur les effets délétères du protoxyde d'azote sur la santé. Alors qu'ils sont bien connus dans d'autres pays, où des morts sont à déplorer, alors que les pouvoirs publics sont alertés depuis plusieurs années, le grand public chez nous demeure encore ignorant ignorant des dangers de ce gaz sur la santé de leurs enfants. Les communiqués de presse ne suffisent plus, l'État doit engager une grande campagne de communication pour informer les Français des risques qu'ils encourent. Sur ce point,

L'interdiction de vente aux mineurs ne réglera pas le problème d'un coup de baguette magique, mais elle sera utile si elle est accompagnée de mesures de prévention. Le délit d'incitation d'un mineur à l'usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs permettra par ailleurs de lutter contre les phénomènes de mode potentiellement dangereux auxquels les jeunes pourraient être exposés aujourd'hui exposés aujourd'hui et à l'avenir. Sur le même modèle que la provocation d'un mineur à la consommation excessive d'alcool, toute personne incitant à l'usage de ce gaz encourra 15 000 euros d'amende, ce qui devrait, espérons-le, en décourager certains. Enfin, je l'ai dit, il est essentiel de renforcer la prévention, par l'information et la communication, au sein des établissements scolaires, sur les risques des conduites addictives en général et pas seulement sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé. Si ces conséquences sont bien réelles et dramatiques, l'addiction elle-même, sous toutes ses formes, doit être appréhendée comme un enjeu de santé publique. On le sait, l'imagination est sans limites lorsqu'il s'agit d'inventer de nouvelles drogues.

Je veux remercier

en effet chaque semaine toujours davantage dans les rues de ma commune, ce qui témoigne de l'utilisation toujours plus importante et toujours plus inquiétante d'un gaz détourné de son usage initial pour ses propriétés euphorisantes et dont on commence à mesurer les effets ravageurs sur la santé. Ce phénomène n'est plus ce seul particularisme local de la métropole lilloise et du département du Nord que certains ont pu évoquer. Il touche aujourd'hui nombre de grandes agglomérations françaises, mais aussi des zones moins denses, comme en attestent les témoignages de nombreux élus rencontrés dans le cadre de la préparation de la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui.

débat et sens. Nous parlons ici d'un gaz utilisé en cuisine dans les siphons à chantilly ou à l'hôpital comme anesthésiant, sauf que personne ne fait de la chantilly ou des opérations à coeur ouvert dans nos rues Le gaz est transféré dans des ballons de baudruche afin d'être inhalé, entraînant alors une euphorie et des rires incontrôlables, certains n'hésitant pas à utiliser plusieurs cartouches dans un seul ballon Alors, me direz-vous, quel problème y a-t-il à se sentir d'humeur joyeuse, voire euphorique ? Chef des urgences du CHRU de Lille et du SAMU, le docteur Patrick Goldstein a pointé du doigt le principal danger de ce gaz, qui « accélère le rythme cardiaque » et « peut avoir des répercussions sur le système neurologique, à savoir le cerveau et la moelle épinière

interdit. Monsieur le secrétaire d'État, prévenir des dangers ne suffit plus. Le moment est venu, je pense, de légiférer pour empêcher autant que faire se peut la propagation du phénomène, notamment chez les plus jeunes, collégiens ou lycéens, pour qui consommer du protoxyde d'azote devient un acte banal, sans aucune conséquence. Pis, chacun voit bien que cette consommation est pour les jeunes la première étape vers d'autres produits stupéfiants, considérant l'absence d'effets du protoxyde pour la santé. Notre proposition de loi, qui, je l'espère, sera adoptée, a pour ambition de préserver autant que faire se peut les mineurs d'un produit pouvant avoir des effets graves sur la santé, ce dont la communauté médicale est plus que persuadée. Préserver les mineurs d'un tel fléau, qui gagne du terrain, c'est le sens du texte. Il a fait l'objet d'aménagements à la suite de son passage en commission.

renforcer l'information sur la dangerosité de l'usage sont autant de mesures sur lesquelles nous ne pouvons que nous accorder pour mettre en place un arsenal permettant d'enrayer cette spirale infernale. Si

de protoxyde d'azote dès leur plus jeune âge et dans l'espace public. Afin d'apporter des réponses concrètes aux alertes des acteurs locaux, des élus, des agents de prévention et des professionnels de la santé, le député Ugo Bernalicis avait déposé au mois de janvier 2019 une proposition de loi pour lutter contre le protoxyde d'azote. Celle-ci fut suivie le 5 avril dernier par une proposition de loi déposée sur l'initiative de Mme Létard et signée par des sénateurs et sénatrices de groupes politiques différents, dont mon collègue Éric Bocquet. Le rapport que l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies a publié au mois de décembre 2018 a relevé une évolution de l'usage et de la consommation du protoxyde d'azote. Jusqu'à présent, c'était uniquement dans les teknivals. Petit à petit, il a fait irruption dans l'espace public.

Face à une telle situation, et devant l'inaction des pouvoirs publics de santé, plusieurs municipalités ont décidé d'en interdire la vente aux mineurs, comme à la Madeleine et à Wattrelos dans le Nord, mais également à Nîmes, à Aulnay-sous-Bois ou à Pont-Sainte-Maxence. La « drogue du pauvre », ainsi qu'on surnomme le protoxyde d'azote, concerne principalement des jeunes impliqués dans le trafic de stupéfiants, les personnes prostituées, les personnes précaires, mais aussi des collégiens et des lycéens, selon le dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues. Aussi, nous ne pouvons rester sans rien faire quand on découvre- c'est le cas à Valenciennes, à Amiens, à Arras ou à Saint-Omer -des centaines de cartouches métalliques de N2O.

est la principale réponse à la consommation du protoxyde d'azote par les mineurs, tandis que le volet préventif est uniquement envisagé par l'apposition d'un pictogramme indiquant l'interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans sur chaque contenant incluant ce produit et avec des actions d'information et de prévention dans les établissements scolaires et l'armée. Les usagers, notamment les plus jeunes, manquent très souvent d'informations sur la dangerosité Des campagnes de prévention et d'information sur le protoxyde d'azote sont donc nécessaires pour limiter les risques. En matière de campagne de prévention, il est fort regrettable que l'agence régionale de santé des Hauts-de-France soit demeurée absente face aux alertes

qui s'accompagne d'une augmentation du nombre de signalements d'effets sanitaires graves, avec atteintes du système nerveux central et de la moelle épinière » et que le Gouvernement accepte de débloquer un fonds d'urgence. Sachant qu'il y a 1,2 million de lycéens et collégiens dans la région des Hauts-de-France, 200 000 euros, c'est 16 centimes d'euro par élève ! Un tel montant est largement insuffisant pour mener une véritable campagne de prévention sur le protoxyde d'azote. Pour nous, ce texte démontre avant tout l'urgence qu'il y a pour le ministère de la santé à prendre des mesures visant à protéger nos enfants et nos jeunes. Les professionnels de santé, qui rencontrent les victimes, sont les premiers à s'opposer aux mesures qui ne seraient que répressives, car elles exposent à un risque de report d'addictions vers d'autres drogues plus fortes et en aucun cas à la diminution de la consommation. Il faut donc développer une politique de prévention et de réduction des risques à l'intention

Ce soutien transpartisan est inhérent au sujet que nous allons étudier. Nous parlons d'une pratique aux conséquences très graves qui touche nos jeunes. Elle est répandue dans les Hauts-de-France, mais aussi dans nombre de grandes villes universitaires.

mais son usage dévié à titre festif à proximité des établissements scolaires fait partie du folklore chez les lycéens et devient même dans les « soirées proto » une tradition chez les étudiants en médecine. Son inhalation procure un effet euphorisant pendant quelques secondes. L'effet est si fugace que les utilisateurs sont poussés à en consommer à répétition, donc à haute dose et à outrance. Ce même gaz est utilisé dans le champ médical coupé avec de l'oxygène, sous le nom de Méopa. Loin de constituer une découverte récente, le protoxyde d'azote fait depuis les années 1800 l'objet d'un double usage, puisqu'il est à la fois anesthésiant et euphorisant. Le Méopa est soumis à une réglementation stricte, qui impose notamment un stockage sécurisé et une déclaration obligatoire en cas de vol. Si le Méopa fait l'objet de contrôle, ce n'est pas le cas du protoxyde d'azote pur. Nos élus sont inquiets : au regard du volume de cartouches vides trouvées sur la voie publique, ils nous ont alertés.

Ce sont des moyens légaux que les maires réclament, afin d'introduire de la teneur dans leurs arrêtés municipaux. Cette proposition de loi est à destination de nos populations, des familles, pour assurer ce devoir de protection des enfants contre ce produit toxique, tout comme nous l'avons fait pour le tabac, l'alcool,

pour un produit unique. Notre rapporteure a modifié le texte initial en commission pour répondre à cette réticence, qui ne peut donc plus nous être opposée. Oui, il y a urgence à légiférer, à informer et à éduquer, parce que les retours de pratique sont là Le rapport de Jocelyne Guidez nous informe que le centre d'addictovigilance de Lille a été saisi à cette date de huit cas graves. Cinq d'entre eux, âgés de 23, 19, 18 et 17 ans, sont atteints de sclérose combinée de la moelle, de neuropathie sensitive et de paraplégie flasque. Ces pathologies sont, dans certains cas, irréversibles. Ce phénomène, connu chez nos voisins britanniques, a provoqué le décès de trente-six personnes depuis 2001. Aux États-Unis, on en dénombre quinze par an. Pour la France, j'évoquerai le cas du jeune Yohan, qui est décédé après absorption de gaz hilarant au mois de décembre 2018 à Lacroix-sur-Meuse. Au sein du groupe Union Centriste, nous estimons qu'il convient d'agir avant que le bilan ne soit plus lourd encore. Il est nécessaire de lutter contre la banalisation et l'incitation à la consommation que nous pouvons constater sur bon nombre de sites internet ou chez des revendeurs classiques. Les cartouches coûtent en magasin rarement plus de 1 euro pièce. Avec la hausse de la demande, un nouveau marché s'est ouvert sur internet, où l'on trouve des bonbonnes à prix cassé, aux allures attrayantes, de surcroît offertes avec des ballons de baudruche, qui permettent l'inhalation en grande quantité et y incitent. En outre, sur Amazon, il est possible d'acheter pour une trentaine d'euros l'équivalent de quatre-vingts cartouches, soit à peine 30 centimes d'euros la dose. Évidemment, une solution consisterait à interdire totalement la vente de ces cartouches. Cependant, Mme la rapporteure l'a évoqué, d'une part, cela serait problématique, puisque ce gaz n'a pas encore trouvé d'équivalent pour son usage domestique et, d'autre part, croyez l'élue du Pas-de-Calais que je suis, interdire dans notre pays n'est pas la bonne solution. Il sera bien facile aux contrevenants de franchir la frontière pour aller se procurer ce produit en Belgique ou aux Pays-Bas, voire de le commander sur internet. C'est à l'échelon européen que nous devons y travailler. En attendant, force est de constater que le dispositif que nous nous apprêtons à adopter apporte une série de solutions pragmatiques et d'application rapide.

deuxième tient à l'interdiction de la vente aux mineurs du protoxyde d'azote, en commerce physique comme en ligne. C'est ce qu'ont fait le Royaume-Uni, certains États américains, Chypre, la Croatie et la Corée.

Les amendements de la commission sont venus opportunément compléter le dispositif initial en élargissant le champ de la proposition de loi à des mesures d'information et de prévention dans le cadre scolaire ou pour la vente en ligne. Devant l'enjeu majeur de santé publique que constitue ce sujet, le groupe Union Centriste votera unanimement en faveur de ce texte, tout en comptant sur la clairvoyance du Gouvernement pour porter ce texte plus loin vers une issue favorable à l'Assemblée nationale. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi de notre collègue Valérie Létard visant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote. dernière intervenante dans la discussion générale, je ne reviendrai pas sur les usages médicaux et culinaires du protoxyde d'azote. Je centrerai mon propos sur ses usages détournés en raison de son effet euphorisant. Ces usages détournés sont observés de manière discontinue depuis 1999. Jusqu'ici, ils se cantonnaient aux milieux festifs alternatifs, tels que les free-parties et les teknivals. À partir de 2015, son usage se répand et se banalise. Il est extrait de bonbonnes industrielles et conditionné dans des ballons de baudruche vendus pour une somme modique de 1 à 2 euros l'unité. Si le protoxyde d'azote est apprécié pour ses effets fugaces et euphorisants, il est aussi utilisé pour potentialiser ou moduler les effets d'autres produits consommés. Facilement accessible sur internet, il est aussi proposé et vendu dans des bars et des établissements de nuit. À partir de 2017, la visibilité du protoxyde d'azote dans l'espace public augmente considérablement. de 2018, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies a publié un rapport soulignant la visibilité du protoxyde d'azote dans l'espace public de la métropole lilloise.

des collégiens et lycéens avides d'expérimentations dans un cadre collectif et « convivial », des jeunes impliqués dans le trafic de drogue et des prostituées qui l'utilisent pour mieux supporter leur condition. L'augmentation de la consommation de protoxyde d'azote semble essentiellement le fait d'une population jeune, voire très jeune. C'est d'autant plus grave que les dangers du gaz ne sont pas suffisamment connus. Plusieurs études ont fait état d'un risque de séquelles neurologiques liées à un usage détourné du gaz pouvant entraîner une atteinte de la moelle épinière- il s'agit là d'une complication grave et peu connue -, mais également des troubles graves du rythme cardiaque pouvant aller jusqu'à la mort. L'intervention du législateur est donc nécessaire. La protection de la population constitue notre priorité. Je pense notamment à la protection des mineurs, qui sont plus vulnérables. La proposition de loi de Valérie Létard vise à interdire la vente de protoxyde d'azote aux mineurs, dans les commerces comme en ligne. Elle punit l'incitation des mineurs à consommer ce gaz et oblige les intermédiaires numériques à en informer leurs abonnés. Son article 2 pénalise l'incitation d'un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs. Il couvre ainsi le protoxyde d'azote et élargit opportunément son champ à d'autres substances. Ce texte contribue à l'information de nos concitoyens en obligeant les industriels à indiquer sur l'emballage la dangerosité du produit et accompagne la politique de prévention menée à l'école. Il a le mérite de présenter un dispositif équilibré, conjuguant protection des mineurs et responsabilisation des industriels face à l'usage détourné du protoxyde d'azote. Mais l'interdiction de la vente aux mineurs ne suffira malheureusement pas. Afin de compléter le travail des sénateurs, je profite de l'examen de cette proposition de loi pour appeler le Gouvernement à lancer une campagne d'information destinée aux usagers,

Nous nous heurtons ici aux limites de ce que peut faire le législateur tant que le protoxyde d'azote n'est pas rangé dans une autre catégorie réglementaire, comme celle des substances dangereuses ou celle des stupéfiants. La commission souhaite avoir l'avis du Gouvernement, afin de savoir ce qu'il est possible de faire pour protéger les jeunes adultes.

en état d'ivresse à consommer du protoxyde d'azote. Par cohérence, notre amendement tend à aggraver les peines prévues par la proposition de loi en cas d'incitation sur mineur en les doublant lorsque la victime est sous l'emprise de l'alcool. objet de pénaliser l'incitation de toute personne en état d'ivresse à consommer du protoxyde d'azote. Ses auteurs cherchent à juste titre à prévenir les mélanges de substances ou l'abus de faiblesse de personnes qui déjà sous l'emprise de l'alcool. Là encore, il s'agit de pénaliser la provocation à faire un certain usage d'un produit légal sans que puisse être invoqué le motif de protection des personnes plus vulnérables

à Mme Valérie Létard. Pour rendre le dispositif opérant, il convient de compléter l'infraction de l'interdiction de vente aux mineurs de protoxyde d'azote en l'assortissant d'une peine d'amende de 3 750 euros. Quel est

Létard. Cet amendement vise à interdire la vente et la distribution de gaz protoxyde d'azote dans les débits de boissons. En effet, on constate une évolution inquiétante du nombre de bars et d'établissements de nuit proposant gratuitement ou à la vente du gaz protoxyde d'azote.

Compte tenu des remarques formulées ce matin en commission des affaires sociales, ce sous-amendement vise à restreindre l'interdiction de vente et de distribution de gaz protoxyde d'azote dans les débits de boissons aux seuls mineurs.

gaz protoxyde d'azote aux seuls débits de boissons. En effet, la rédaction actuelle de l'amendement n° 1 rectifié étend cette interdiction aux commerces de détail alimentaires.

englobe aussi bien les supermarchés où se vendent également les cartouches de gaz à usage culinaire. Une telle interdiction quasiment générale risquerait de rendre disproportionnés les moyens retenus par ce texte pour atteindre l'objectif de santé publique fixé et donc de se heurter au droit européen. Le sous-amendement n° 8 a pour objet de ramener l'interdiction de vente aux seuls mineurs dans les lieux de vente de boissons alcoolisées. Sa rédaction est plus ambigüe, mais son esprit est en tout cas satisfait par le texte, qui interdit la vente de protoxyde d'azote aux mineurs dans tous commerces ou lieux publics. au sous-amendement n° 7, il vise à restreindre l'interdiction de vente aux lieux de consommation d'alcool. Tel qu'il est rédigé, il est sans doute trop imprécis pour être opérant. Sans doute pourrait-on viser les débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique, mais, là encore, l'interdiction de vente d'un produit restant légal risque de revêtir un caractère trop général

et de l'amendement visant à interdire la vente et la distribution de gaz protoxyde d'azote dans les débits de boissons.

également de notifier le plus rapidement possible à la Commission européenne ses futures dispositions, comme nous y oblige la directive européenne 2015/1535, que le texte puisse entrer en vigueur dans les prochains mois. Une vive réactivité contribuera à une efficacité salvatrice. Mes chers collègues, nous faisons face à un enjeu social et à un problème de santé publique. Songez que le protoxyde d'azote, dans son usage médical, est mélangé

rester avec nous. Il m'a donc demandé de me substituer à lui, ce que je fais bien volontiers : le grand-père que je suis est évidemment extrêmement sensible à ce genre de législation. Il y a une urgence extrême

devons faire la démarche nous-mêmes à l'Assemblée nationale, pour faire en sorte que le texte soit adopté le plus rapidement possible. Si Valérie Létard y consent, je l'aiderai

La séance est reprise. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution,

-à la nomination de M. Bertrand Munch aux fonctions de directeur général de l'Office national des forêts. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2020

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avoir un débat sur la politique énergétique de la France et sur la place de ce fleuron national qu'est EDF, c'est aborder simultanément des sujets de politique industrielle, de sécurité nationale, de transition énergétique et de protection de l'environnement. À nos yeux, la politique énergétique d'une nation constitue l'une des principales politiques publiques transversales qu'un pays doit mener. Or, depuis plus de deux ans, il est difficile d'identifier celle que porte le Gouvernement. C'est pourquoi nous avons décidé d'inscrire ce débat dans le cadre de l'espace réservé de notre groupe. donnera l'occasion de vous interroger, et il vous permettra, je l'espère, de clarifier les ambitions du Gouvernement. L'équation à résoudre est complexe. Définir une politique énergétique, c'est fixer des priorités entre différents enjeux parfois contradictoires. Les principaux enjeux

viser notre indépendance énergétique ; garantir la production et l'acheminement de l'énergie en toutes circonstances ; choisir des sources de production sûres pour la population et pour l'environnement ; enfin, préserver la qualité de nos paysages. Tous ces objectifs sont louables, mais difficilement conciliables. Vous devez faire des choix, établir une hiérarchie des priorités. Après le premier choc pétrolier, l'indépendance énergétique, avec le nucléaire, et la maîtrise du coût pour le consommateur final ont prévalu, et ce quasiment jusqu'à aujourd'hui. L'entreprise nationale était alors le bras armé de la Nation pour mettre en oeuvre cette politique. L'État lui fixait ses priorités. Aujourd'hui, nous sentons un flottement dans la stratégie, qui se répercute sur EDF, désormais confrontée, de surcroît, à des entreprises concurrentes sur le plan international. Nous ne savons plus si EDF répond à la politique choisie par le Gouvernement ou si elle agit en entreprise indépendante, alors que l'État en détient encore 83 %. Il est temps de définir le positionnement des représentants de l'État au sein du conseil d'administration d'EDF et de clarifier les buts visés dans les domaines suivants quel degré de volontarisme dans la stratégie de décarbonation et quel mix énergétique ? Quel avenir pour la filière nucléaire ? Quelle politique de prix, eu égard à la compétitivité de notre économie et à la maîtrise des charges pour les consommateurs ? s'agisse de la décarbonation ou du choix des sources de production d'énergie, le lien entre l'État et EDF n'est pas clarifié, et les décisions successives ne reflètent pas de vision stratégique. Il faut lever les confusions en matière de mix énergétique et affirmer la position française. Le précédent gouvernement a imposé à EDF la fermeture de la centrale de Fessenheim, contre toute logique de sûreté ou financière. Le gouvernement auquel vous appartenez a fait le choix d'éteindre les quatre centrales à charbon. Il y a quelques semaines, le P-DG d'EDF, M. Lévy, annonçait la construction souhaitable de six nouveaux réacteurs nucléaires en France de type EPR, alors même que celui de Flamanville a déjà pris onze ans de retard et que son coût a triplé Le Président de la République annonçait en 2018 la fermeture de quatorze réacteurs à l'horizon de 2035, sans préciser les éventuelles nouvelles constructions. Dans le même temps, vous avez souhaité, à juste titre, développer des sources d'énergies décarbonées. Cet enchaînement et même ces contradictions, au moins apparentes, nuisent à la compréhension pour les parlementaires que nous sommes, mais aussi pour les salariés d'EDF. Vous avez souhaité diminuer la part du nucléaire dans le mix énergétique à hauteur de 50 % à l'horizon de 2035. Force est de constater que, pour remplacer plus de 20 % de la production par des énergies renouvelables, sans compter les hausses de consommation à venir, il faudra un engagement plus fort dans le développement des énergies solaire, éolienne, hydraulique ou encore géothermique. impliquera plus de moyens, plus de volontarisme et surtout plus d'acceptation de la part des citoyens. Elle doit aussi engendrer plus de mesures d'économies d'énergie. Quand allons-nous réellement progresser en matière d'énergie renouvelable ? Notre pays a par exemple, sans doute, le meilleur « terrain de jeu » pour le développement de l'éolien en mer. Nous restons malheureusement des nains mondiaux en la matière. En matière d'éolien terrestre, nous observons une schizophrénie bien française : on alterne entre volonté de développer une énergie propre et refus de la voir s'installer sur son territoire. Ce manque d'acceptation de la part des habitants illustre parfaitement un syndrome assez répandu : le « pas dans mon jardin », en bon français. Pourtant, il faudra parfois faire des choix entre la préservation des paysages et le développement des modes de production renouvelables. Comment dépasser certains blocages ? Peut-être en présentant le coût complet, financier et environnemental, des différentes sources d'énergie. En outre, la production locale, voire l'autoproduction sont des thématiques qui se développent. Quel équilibre voyez-vous entre ce type de ressources et les grandes productions nationales ? Augmenter le nombre de points de création d'énergie peut rapprocher la production des territoires, voire leur assurer une certaine autonomie, mais nécessite des compromis, notamment environnementaux. Le deuxième positionnement que l'on pourrait attendre du Gouvernement vis-à-vis d'EDF concerne l'avenir de la filière nucléaire. Avec cinquante-huit réacteurs, la France produisait en 2017 près des trois quarts de son électricité grâce au nucléaire. À titre de comparaison, aux États-Unis, seulement 20 % de l'électricité provient du nucléaire, contre 11,6 % en Allemagne et 4 % en Chine. Ces chiffres résultent des choix forts et ambitieux, depuis soixante-dix ans, d'une forme de stratégie gaullienne de souveraineté énergétique. L'énergie d'origine nucléaire nous permet par ailleurs de produire peu de gaz à effet de serre. Nous estimons qu'il est important de conserver notre spécificité pour atteindre les objectifs fixés dans l'accord de Paris. Je le disais plus tôt, les annonces en matière de nucléaire sont contradictoires et les choix du passé pèsent sur la santé d'EDF. Aujourd'hui, le nucléaire français vacille, fragilisé par le poids de la dette et par le montant exceptionnel des investissements nécessaires pour rénover le parc et les nombreux retards de chantier retards sur l'EPR de Flamanville et sur l'EPR finlandais, risques pesant sur les investissements et la rentabilité du projet d'Hinkley Point. Tout cela pèse sur notre électricien, aujourd'hui endetté à près de 37 milliards d'euros- ce montant dépasse même le double si l'on y ajoute les emprunts obligataires -, soit trois fois plus qu'il y a dix ans, sans compter les investissements obligatoires, comme celui du grand carénage, qui devrait atteindre 100 milliards d'euros d'ici à 2030. Outre la mauvaise santé financière d'EDF, dont son actionnaire ultra-majoritaire ne peut se désintéresser, vous devez forcément garder à l'esprit une préoccupation humaine et technique : il s'agit d'associer les salariés et les agents, de les motiver et de mettre en avant leurs savoir-faire. Il faut accompagner ces changements, y compris pour préserver les connaissances technologiques nécessaires pour préparer l'avenir. Il ne faut pas non plus, pour sauver les apparences, démanteler et séparer les activités d'EDF, comme le projet Hercule pourrait le laisser penser. Le troisième et dernier positionnement stratégique que je souhaite aborder a trait au prix de l'énergie.

l'un des rares avantages comparatifs dont bénéficient nos entreprises. La hausse des prix de gros sur les marchés de l'électricité a conduit les fournisseurs alternatifs à se reporter sur l'Arenh. Le débat autour de cet accès régulé a eu lieu lors de l'examen du projet de On pressent que ce modèle atteint ses limites. EDF continue d'investir et prend des risques, tandis que ses concurrents alternatifs font des choix d'opportunité entre le marché mondial et le marché protégé. Ce modèle amortit les hausses pour le consommateur final, mais ne reflète pas le véritable coût de l'électricité. Face à la crise des « gilets jaunes » et aux demandes en matière de pouvoir d'achat, M. le Premier ministre annonçait, en décembre 2018, le gel des tarifs de l'électricité et du gaz jusqu'en mai 2019. mesure n'a pas empêché une hausse en juin 2019, la plus forte depuis la libéralisation du marché en 2007, suivie d'une autre au mois d'août, due à l'augmentation des coûts de distribution. Plusieurs questions se posent donc désormais. Quelle est la stratégie du Gouvernement en matière de prix de l'électricité ? Faut-il faire payer le prix réel au consommateur ? Allez-vous revoir le rapport entre EDF et ses concurrents, qui fait peser sur la seule entreprise historique le coût moindre de l'énergie en France ?

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, le débat qui nous rassemble cet après-midi est au coeur de la réponse à l'urgence climatique, et le défi est de taille : changer notre production et notre consommation d'énergie, c'est changer plus de cinquante ans d'habitudes à tous les niveaux. Relever ce défi, c'est d'abord une question de visibilité, de cap. C'est pour cela que la loi Énergie-climat nous donne un objectif clair : la neutralité carbone en 2050. C'est donc une politique de transition énergétique que nous devons mettre en oeuvre. Cela implique d'abord de sortir des énergies fossiles et de commencer par tourner la page du charbon. C'est pourquoi, avant 2022, nous allons fermer les quatre dernières centrales qui utilisent encore cette ressource. Ces fermetures peuvent aussi être une occasion d'innover : à Cordemais, EDF mène un projet de production de biomasse à partir de déchets de bois, qui commencerait sa production en 2022. Ce dispositif alimenterait la centrale électrique de manière transitoire avant d'alimenter des réseaux de chaleur.

Là encore, notre cap est clair, avec un objectif intermédiaire : baisser ces consommations de 20 % d'ici à 2030. Bien sûr, tous les secteurs sont concernés par cet effort. Toutefois, cet après-midi, je pense principalement à deux domaines, que vous connaissez bien pour en avoir longuement débattu ces derniers mois.

Sur les dix ans de la PPE, nous devons baisser les consommations du secteur d'environ 15 % et multiplier les nouveaux vecteurs énergétiques, l'électricité, bien sûr, mais aussi l'hydrogène. Le second levier de la sobriété énergétique, c'est le bâtiment, qui représente près de la moitié de la consommation énergétique. Vous avez voté la fin des passoires thermiques : il nous faut maintenant la mettre en oeuvre. Eh oui ! Tout en rénovant l'existant, nous devons veiller à minimiser la consommation énergétique des nouveaux bâtiments, car les constructions d'aujourd'hui seront debout à la fin du siècle. C'est donc dès le départ qu'il nous faut garantir les économies d'énergie. 2020, ou RE 2020, sera l'occasion de mettre en oeuvre cette nouvelle ambition. La maîtrise des consommations énergétiques en complément de tarifs maîtrisés est un enjeu essentiel pour que la transition énergétique ne laisse aucun Français sur le bord de la route. Une politique énergétique visant la neutralité carbone au milieu du siècle, c'est aussi la massification des énergies renouvelables. Nous avons un rendez-vous en cours de route : 33 % d'ENR dès 2030.

outre, 40 % de l'électricité sera produite à base d'ENR. À ce titre, les deux filières ayant le plus fort potentiel sont connues : l'éolien et le photovoltaïque. à l'éolien en mer depuis 2012. Pour exploiter pleinement ce potentiel, nous visons à présent l'attribution d'un gigawatt offshore chaque année d'ici à 2024. ce qui concerne le photovoltaïque, notre objectif est de multiplier par cinq la puissance installée d'ici à 2028 pour atteindre plus de 36 gigawatts. Parce que les objectifs demandent aussi des moyens, au total, sur la décennie, 30 milliards d'euros seront mobilisés pour le développement des ENR électriques. Cette politique volontariste s'accompagne d'un objectif de diversification du mix électrique : nous allons réduire la part du nucléaire à 50 % à l'horizon de 2035. Je suis convaincue que cette diversification des sources rendra notre système plus résilient ; dans cette politique énergétique vers la neutralité carbone, EDF a tous les atouts. mentionné la baisse de la part du nucléaire en 2035. Pour EDF, cela signifie concrètement fermer quatorze réacteurs. Il s'agit d'une transition majeure, que nous allons accompagner, pour les salariés, les territoires et l'entreprise. La fermeture des deux réacteurs de Fessenheim dès l'année prochaine sera l'occasion de le démontrer. Au-delà, quels que soient les choix du mix énergétique de la France pour le milieu du siècle, EDF sera l'une des clés de voûte. EDF sera tout d'abord présente à travers les réseaux. Ces éléments centraux de notre système électrique nécessiteront des adaptations et des investissements importants dans les prochaines années, avec une production plus décentralisée, raccordée sur les réseaux de distribution ou les nouveaux parcs d'éolien offshore sur le réseau de transport ; avec les nouveaux usages, tels que la mobilité électrique ; avec une flexibilité plus importante des moyens de production et de consommation. Enedis et RTE joueront donc un rôle central pour accompagner la transition de notre système électrique. S'agissant du mix énergétique, notre approche doit être raisonnée. étudier tous les scénarios, en détailler les avantages et les inconvénients pour prendre une décision éclairée. En effet, cette transition énergétique pose des questions qui engagent notre pays tout entier. Peut-on avoir un système 100 % renouvelable, et à quel coût ? Dans quelles conditions la filière nucléaire pourrait-elle déployer un nouveau programme ? Et que ferons-nous des déchets ? Si le choix se porte sur un nouveau programme nucléaire, EDF sera évidemment au premier plan. Elle devra être le fer de lance de la filière. Si l'on choisit de se tourner davantage vers l'énergie renouvelable, EDF est déjà au rendez-vous. Parmi ses projets, on compte quatre des sept parcs éoliens en mer et 30 gigawatts de photovoltaïque annoncés d'ici à 2035. Mesdames, messieurs les sénateurs, oui, la transition énergétique de la France est un défi mais ce défi, nous allons le relever avec les acteurs historiques de l'énergie en France. Je suis convaincue qu'EDF en a les moyens et qu'ensemble nous y arriverons ! Nous allons maintenant Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

renouvellement des concessions nationales. Ainsi, le département des Pyrénées-Atlantiques est concerné par le renouvellement des trois concessions hydroélectriques de la vallée d'Ossau, située en Béarn, près de Pau. Ces délégations de service public de l'État sont arrivées à leur terme le 31 décembre 2012. Depuis, elles n'ont pas été renouvelées. S'ensuit une situation juridique instable de délais glissants, prorogeant de fait les concessions aux conditions antérieures.

Comme vous le savez, la carence de l'État en la matière est susceptible d'engager sa responsabilité, tant en droit interne que du point de vue du droit européen. risque également de devoir acquitter des indemnités importantes, compte tenu des dépassements de délais constatés. Désormais, il est donc plus qu'urgent que l'État engage les démarches visant à mettre fin à la situation actuelle, non conforme au droit, de prorogation tacite des concessions. Pour ce faire, plusieurs solutions existent. Elles vont du lancement d'une nouvelle procédure de délégation de service public

Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la formule que l'État retiendra, le traitement rapide de cette situation s'impose. Il faut conclure, chère collègue ! Qu'envisage de faire l'État sur ce sujet : se mettre en phase avec le droit européen

est à Mme la ministre. Le Gouvernement soutient pleinement l'hydroélectricité : c'est une énergie flexible et compétitive. En outre, les ouvrages d'hydroélectricité présentent des enjeux majeurs, qu'ils soient sociaux, économiques, d'aménagement du territoire, de sûreté ou de partage de la ressource en eau. suite des deux mises en demeure formulées par la Commission européenne, en octobre 2015 au plan concurrentiel et en mars 2019 quant au respect des droits des concessions,

Ces échanges n'ont pas abouti à une solution satisfaisant les deux parties. Le droit communautaire ne permet pas d'envisager l'option que vous présentez, madame la sénatrice, de prolongation des contrats de concession contre travaux. À côté de l'option de mise en concurrence, le Gouvernement explore actuellement avec la Commission européenne une nouvelle voie permise par le droit des concessions : une quasi-régie permettant d'octroyer sans mise en concurrence des concessions à une structure publique dédiée. aucune décision n'est prise à ce stade : les discussions se poursuivent avec la Commission européenne. Le renouvellement des concessions, par le biais d'une mise en concurrence ou une structure publique dédiée, est une politique que nous souhaitons mener pour optimiser la gestion de nos barrages et y relancer l'investissement, tout en redistribuant des ressources financières vers les territoires par de nouvelles redevances. En attendant qu'une solution structurelle soit mise en oeuvre, nous avons mis en place en juin 2019 une redevance sur les concessions en délais glissants. Cette dernière, égale à 40 % du résultat des concessions échues, est reversée aux collectivités. Elle peut donc répondre aux difficultés financières que vous évoquez. La parole est à M. Gérard Longuet. L'accès

est à Mme la ministre. La discussion engagée avec la Commission européenne porte bien sur la régulation du nucléaire historique. D'ailleurs, pour un nouveau projet de production d'électricité, qu'il soit nucléaire ou renouvelable, il n'y a pas de

au prix du carbone ou encore aux crises que connaissent les pays producteurs de pétrole. C'est dans cet esprit que nous poursuivons nos discussions avec la Commission, pour sécuriser dans la durée la régulation du nucléaire historique.

accepte une bonne fois pour toutes que le droit de la concurrence ne doit pas priver l'Europe d'atouts industriels majeurs, à l'instar du nucléaire d'EDF.

à l'aune du défi climatique. Pour ce faire, il faut commencer par éviter la mort cérébrale de l'Europe de l'énergie, qui doit articuler sécurité énergétique et priorité climatique. En France, nous devons relever l'ambition de nos politiques publiques et changer de braquet, à toutes les échelles. Il s'agit d'un véritable effort de guerre

d'abord savoir ce qui est « vert » et ce qui ne l'est pas. La taxonomie peut, en apportant la clarté nécessaire, permettre de lutter contre l'éco-blanchiment. Madame la ministre, le nucléaire, énergie décarbonée, doit-il être maintenu dans la taxonomie européenne ?

la mise en concurrence des concessions hydroélectriques conduira à la désoptimisation de la production de ces outils. Madame la ministre, vous avez indiqué en commission vouloir trouver un chemin pour éviter cette hérésie : où en est-on ? Enfin, la stratégie industrielle en faveur de la transition ne doit pas se construire construire façon puzzle. Ainsi, à EDF, nous avons besoin d'un projet industriel, et non d'un projet de scission de type Hercule. Chez Engie, confirmez-vous que l'État valide l'orientation du conseil d'administration consistant à vendre les infrastructures gazières, qui pourtant participent à notre souveraineté énergétique ?

Nous avons des objectifs et un cadre actualisé l'année dernière ; des législations ont été adoptées en 2018 et 2019,

ETS. Nous plaidons pour la fixation d'un prix minimal du carbone à l'échelle européenne et pour la mise en place d'un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, pour que nos industriels, qui paient un prix du carbone carbone appelé à augmenter, ne soient pas pénalisés par rapport aux industriels de pays moins engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique. S'agissant de la taxonomie, les discussions sont en cours ; elles ont été abordées aujourd'hui et le seront de nouveau la semaine prochaine.

J'aurais bien aimé, madame la ministre, vous entendre sur le projet Hercule et la décision du conseil d'administration d'Engie de vendre certaines infrastructures gazières.

qui contribuent à optimiser les infrastructures et, partant, nous permettent d'envisager l'avenir de manière positive. Un des principaux défis auxquels nous devons répondre est l'augmentation de la flexibilité de notre système électrique pour mieux répondre aux pics de consommation. Une technologie le permet : les stations de transfert d'énergie par pompage. Or, actuellement, nous n'en avons aucune dans les Pyrénées, même si un projet est à l'étude sur le site d'Orlu, en Ariège.

importante à la fois pour le système électrique national, pour l'atteinte de nos objectifs d'énergies renouvelables et pour le développement économique local. Le maintien et le développement de cette ressource dans le respect des enjeux environnementaux sont indispensables pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques ambitieux que nous nous sommes fixés. Si la production hydroélectrique peut connaître des fluctuations d'une année à l'autre en fonction de l'hydraulicité, la puissance installée en France métropolitaine continue de progresser ; elle est actuellement de 25,5 gigawatts. Le potentiel restant est limité par le taux d'équipement, déjà élevé, et par les enjeux de protection de l'environnement, mais il existe encore une marge de progression et d'optimisation du parc. Dans ce cadre, le Gouvernement soutient la réalisation de nouveaux investissements pour développer l'hydroélectricité, dans le respect, naturellement, des objectifs de bon état de la ressource en eau et de reconquête de la biodiversité. À la faveur du projet de révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie,

Il est prévu que cet objectif soit atteint, essentiellement, par des optimisations ou des équipements complémentaires sur les barrages existants et, dans une moindre mesure, par quelques nouveaux sites, de puissance limitée dont le développement serait compatible avec les objectifs de biodiversité. Le projet de PPE identifie également un objectif de développement des stations de transfert d'énergie par pompage, les STEP.

sur l'élaboration d'un scénario « 100 % renouvelable ». Cette démarche est un signe fort de l'ambition écologique du Gouvernement elle montre que l'inscription dans la loi Énergie-climat d'objectifs tels que la réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production d'électricité ne saurait constituer une fin en soi ni empêcher toute réflexion sur la généralisation des énergies renouvelables. Vous avez expliqué que l'arbitrage entre le « 100 % renouvelable » et la construction de nouvelles centrales nucléaires pourrait être précisé à partir de 2021. pouvez-vous nous renseigner sur les éléments qui seront déterminants dans cet arbitrage ? En particulier, la mise en service de l'EPR de Flamanville constituera-t-elle un facteur essentiel dans la prise de décision ? outre, comment le groupe EDF pourrait-il être associé, le cas échéant, à la définition et à la mise en oeuvre du « 100 % renouvelable

et tous les scénarios, depuis la construction de nouveaux réacteurs nucléaires jusqu'à la poursuite d'un mix 100 % renouvelable. Plusieurs sujets sont actuellement à l'étude, qui nourriront la prise de décision du Gouvernement. Je pense en particulier

la capacité de la filière nucléaire à relever, sur les plans de la qualité industrielle et de la maîtrise des délais, le défi que représenterait la relance de la construction de réacteurs dans des délais et des coûts impartis, aux modalités de gestion des déchets produits par un nouveau parc, si la aux conditions de financement d'un tel programme de construction. Bien sûr, je pense aussi,, à la faisabilité technique et économique d'un système électrique fondé à 100 % sur des énergies renouvelables. dernier scénario, nous avons, il est vrai, lancé une étude avec l'Agence internationale de l'énergie et RTE. Ce travail nous permettra de comparer plusieurs options de mix électrique dans tous leurs aspects : faisabilité, sécurité d'approvisionnement, coûts,

La parole est à Mme la ministre.

il est demandé de jouer un rôle central dans la transition écologique du pays : d'une part, en poursuivant l'exploitation du parc nucléaire existant jusqu'à cinquante ans et, d'autre part, en développant massivement les énergies renouvelables, le stockage et les réseaux intelligents. Dans ce contexte, nous avons demandé au président d'EDF de nous faire des propositions d'évolution de l'organisation du groupe pour répondre au mieux à ces enjeux. C'est un sujet sur lequel l'entreprise travaille et qui, naturellement, doit faire l'objet de concertations avec les partenaires sociaux. La priorité du Gouvernement est que l'entreprise dispose de capacités d'investissement accrues pour participer pleinement à la transition énergétique dans ses différentes composantes- nucléaire, réseaux, énergies renouvelables, services énergétiques. C'est dans ce cadre que la réflexion est engagée

d'éviter la mise en concurrence dans le cadre de la directive Concessions. S'agissant des énergies marines, je suis vraiment très confiante sur le potentiel

Le projet auquel nous pensons dans les Hauts-de-France n'est pas situé dans un estuaire : il s'agirait de construire une gigantesque digue en mer, présentant d'autres avantages.

Leur inquiétude ne portait pas encore sur le régime de retraite, mais sur l'avenir de leur métier et, plus largement, de l'entreprise historique EDF.

Pourtant, l'arrivée à échéance des concessions et le souhait de Bruxelles de les voir mises en concurrence inquiètent EDF et ses salariés, mais aussi les collectivités territoriales. Dans cette période d'incertitude, EDF continue à investir, mais, à mon avis, de façon trop mesurée. Cette menace de mise en concurrence et de perte des concessions se traduit par un manque à gagner pour EDF, par des investissements français qui risquent d'être perdus,

indispensable à notre système électrique, à l'atteinte de nos objectifs de développement des énergies renouvelables et au développement économique de nos territoires. Aujourd'hui, le droit français prévoit, en conformité avec le droit européen, que les concessions hydrauliques échues doivent être renouvelées par mise en concurrence. Plusieurs concessions hydroélectriques sont déjà arrivées à échéance depuis la fin de 2011, sans que la procédure concurrentielle soit engagée. Compte tenu des enjeux sociaux, économiques et écologiques liés à l'hydroélectricité, les gouvernements successifs se sont, disons, donné le temps de réfléchir

une lourde responsabilité dans la casse de cet outil, qui s'est révélé être un cheval de Troie masquant, d'ailleurs mal, une priorité de rendement.

Pour dégager ces ressources, il faut s'appuyer à la fois sur des financements publics et sur des financements privés. S'agissant des financements publics, nous avons considéré qu'il était important de donner davantage de lisibilité aux financements mobilisés en faveur du climat. C'est le sens de la démarche de ,qui permet

le défi financier posé par sa dette, les besoins de financement des investissements et le maintien injustifié de l'Arenh ; le défi de la souveraineté énergétique nationale, l'État et les collectivités territoriales devant garder la totale maîtrise de la gestion de ce bien premier et stratégique qu'est l'électricité. Pour répondre à ces objectifs dans l'intérêt général de la Nation, deux conceptions s'opposent : celle du Gouvernement, exprimée dès mars 2016 à l'Assemblée nationale par le Président de la République, qui était alors ministre de l'économie, à savoir la scission des composantes du groupe, du démantèlement- c'est le mot qu'il a employé lui-même ce jour-là-, à l'instar de ce qui s'est passé et se passe encore pour Engie, ex-Gaz de France ; l'autre conception est celle de ceux qui pensent comme moi que l'intégration actuelle du groupe EDF est un atout majeur et qu'elle doit être confortée, non par dogme, mais par souci d'efficacité à long terme pour une industrie de réseaux par nature très capitalistique, dans l'intérêt premier des clients et des collectivités locales, qui doutent et craignent la remise en question du régime des concessions et des principes qui ont fait preuve de leur efficience, comme celui de la péréquation tarifaire. Madame la ministre, dans ce contexte flou, anxiogène pour les personnels concernés, attisé en particulier par l'hypothèse que vous avez exprimée d'un mix électrique à 100 % de ressources renouvelables, pouvez-vous préciser l'épure et la justification par le Gouvernement du projet Hercule que vous avez soumis au président d'EDF ?

qui propose des projets de réorganisation d'EDF. Le Gouvernement pose un cadre pour la politique énergétique- il me semble que c'est son rôle-, et il souhaite qu'EDF trouve la meilleure organisation, dans le cadre d'une entreprise intégrée,

dans ce défi de la transition énergétique. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, il est demandé à EDF à la fois de poursuivre l'exploitation du parc nucléaire existant jusqu'à cinquante ans et de participer à un développement massif des énergies renouvelables. Je pense qu'EDF répond bien à ces différents défis,

vrai ! Permettez-moi de souligner l'enjeu majeur que constitue pour nous la maîtrise totale des réseaux. Après vous avoir entendue, on ne sait toujours pas comment Enedis pourrait rester totalement publique, par exemple en étant intégrée dans l'entité EDF Vert, dont le capital sera ou serait privatisé.

Sur le plan énergétique, elle est garante de notre indépendance et le fer de lance de notre transition. Sans l'engagement résolu de notre grand énergéticien, l'objectif de neutralité carbone découlant de la loi Énergie-climat ne pourrait être atteint. Or EDF est actuellement confrontée à de lourdes difficultés. Le groupe fait face au mur de l'investissement : grevé d'une dette de 33,4 milliards d'euros, il doit parvenir à financer le grand carénage, les EPR de Flamanville et d'Hinkley Point, les plans solaire et stockage, sans compter les six nouveaux projets d'EPR à l'étude.

sont symptomatiques de ces difficultés. Sans l'appui de l'État, le plan d'action que doit présenter EDF sur ce dossier sera bien impuissant pour sortir de l'ornière. Le projet de réorganisation Hercule est présenté comme le moyen de dégager des capacités d'investissement supplémentaires, mais ce serait au prix de l'ouverture du capital d'un

privilégier depuis plusieurs années la perception des dividendes sous forme d'actions pour laisser des marges de manoeuvre financières à l'entreprise. Notre

figure la nécessité de disposer d'une énergie, certes décarbonée, mais aussi compétitive et surtout disponible, notamment pour faire face aux heures de pointe et aux variations saisonnières. De même, la nécessité d'assurer la souveraineté énergétique de notre pays a été régulièrement soulignée comme un élément stratégique. Le séisme qui a frappé l'Ardèche en novembre dernier a entraîné l'arrêt par précaution de trois réacteurs nucléaires. La puissance nucléaire française est ainsi tombée à 40 gigawatts du fait de l'arrêt pour maintenance d'autres réacteurs. Aussi nous sommes-nous retrouvés dans la configuration prévue à l'horizon de 2035 en termes de puissance nucléaire disponible. Durant cette période, les vents étaient faibles et l'ensoleillement limité. Pour faire face à la demande énergétique, les centrales fonctionnant au charbon, au gaz ou au fioul ont donc tourné à plein régime. La France, qui était quelques jours auparavant exportatrice d'électricité, est devenue importatrice, essentiellement depuis l'Allemagne et l'Espagne. Mes questions sont donc les suivantes : n'y a-t-il pas un risque pour la France de voir croître sa dépendance aux importations dans un contexte où beaucoup de pays européens prévoient eux aussi de fermer des centrales au fioul ou au charbon produisant à la demande- on comprend pourquoi sur le plan environnemental -, cela en espérant qu'un pays voisin puisse, en cas d'absolue nécessité, leur fournir l'électricité dont ils ont besoin ? La souveraineté de notre pays a-t-elle été appréhendée dans la PPE sur le moyen terme ? N'y a-t-il pas nécessité de se doter d'une véritable stratégie européenne coordonnée pour anticiper les situations de crise ? La parole est à Mme la ministre. Le début

: plusieurs réacteurs ont été mis à l'arrêt par précaution et d'autres étaient encore en cours de maintenance, ce qui a porté notre capacité nucléaire à 40 gigawatts sur les 63 gigawatts installés.

Cet épisode interroge indéniablement notre souveraineté énergétique et notre dépendance aux pays voisins. Il met aussi en lumière la nécessité de diversifier le mix électrique français pour le rendre plus résilient à des événements exogènes et, donc, moins dépendant de la production d'origine nucléaire. Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit un développement extrêmement volontariste des capacités de production d'énergies renouvelables, mais également des dispositifs permettant d'accroître la flexibilité de notre système électrique, notamment ses capacités d'effacement ou de stockage, par exemple sous forme de STEP. Il s'agit notamment de disposer d'une capacité de production de 74 gigawatts, soit une augmentation de 50 % par rapport à la capacité actuelle, et entre 102 et 103 gigawatts en 2028, soit un doublement. Il s'agit aussi d'augmenter nos capacités d'effacement pour les porter à 6,5 gigawatts. Le projet de programmation pluriannuelle

EDF est le premier producteur européen d'électricité, mais cette entreprise doit gérer à l'heure actuelle une montagne de dettes récemment estimées à 37 milliards d'euros. Les inquiétudes se multiplient au regard des 46 milliards d'euros que représente le coût de construction de six nouveaux réacteurs nucléaires. Le coût de construction d'un réacteur,

Le scénario 100 % énergies renouvelables est en train de s'écrire aux dépens de l'électricien national surendetté, dont les choix stratégiques semblent de plus en plus soumis aux aléas de la politique. La dette d'EDF pèse, à tous égards et à court ou moyen terme, directement sur les Français. C'est pourquoi le Gouvernement a demandé à Jean-Bernard Lévy de remettre un projet de réorganisation de l'entreprise nommé Hercule. Ce projet d'envergure semble susciter un mécontentement général au sein de l'entreprise, que ce soit des salariés, des syndicats ou de la direction. En effet, cette réorganisation de l'entreprise vise à diviser la société en deux entités, en séparant les activités de production d'électricité et celles de vente et de distribution. Deux entreprises distinctes seraient alors créées : d'un côté, un « EDF Bleu », nationalisé, regroupant le nucléaire et l'hydraulique, lourdement endetté et à la charge exclusive de la collectivité ; de l'autre, un « EDF Vert », qui chapeauterait les énergies renouvelables, le commerce, Enedis et le réseau des petites lignes électriques et serait ouvert aux investisseurs privés. Un projet de réorganisation d'EDF semble inévitable pour sauver l'entreprise, ... Il faut conclure, cher collègue ! ... mais il est à la peine. Madame la ministre, pourriez-vous nous éclairer sur les actions du Gouvernement pour sauver cette entreprise publique et les avancées de ce projet ? La parole est à Mme la ministre. La dette

EDF a mené des actions structurantes depuis plusieurs années pour assurer la maîtrise de sa trajectoire financière. De son côté, l'État a apporté un concours substantiel au groupe EDF au cours des dernières années, notamment au travers de la recapitalisation menée

le Gouvernement demande à EDF de jouer un rôle central, d'une part, par la poursuite de l'exploitation du parc nucléaire existant jusqu'à cinquante ans et, d'autre part, par le développement massif des énergies renouvelables, du stockage et des réseaux intelligents. Je note avec satisfaction qu'EDF prend toute sa place dans le développement de nos énergies renouvelables. Par exemple, quatre des sept parcs éoliens offshore ont été attribués à EDF. C'est dans ce contexte que le Gouvernement a demandé au président d'EDF de réfléchir à l'évolution de l'organisation du groupe,

une discussion est engagée avec la Commission européenne sur la sécurisation de la régulation du nucléaire historique. Une telle régulation est nécessaire pour donner de la visibilité à l'entreprise

Je m'interroge sur la décision d'arrêter les études préalables à la réalisation du prototype Astrid, réacteur à neutrons rapides de quatrième génération. La mise au placard de ce projet a en effet suscité beaucoup de réactions négatives, notamment au sein de la filière nucléaire française. La France a longtemps été aux avant-postes du développement de cette filière de surgénérateurs. Les caractéristiques de ces réacteurs apparaissent particulièrement adaptées à la situation énergétique et environnementale, qui se dessine à la fois pour notre pays et pour la planète. ont un rendement infiniment plus élevé que les réacteurs actuels : avec la même quantité d'uranium, ils produisent de soixante à cent fois plus d'électricité. De plus, tout comme les réacteurs nucléaires actuels, ces réacteurs de quatrième génération produiraient de l'électricité sans émettre de gaz à effet de serre. Ils permettraient également le recyclage complet des matières énergétiques et la transmutation de certains types de déchets nucléaires à longue durée de vie. C'est une forme d'économie circulaire tant souhaitée par nos concitoyens et une partie de la réponse à la problématique du stockage des déchets.

L'électricité nucléaire est nécessaire au mix énergétique. Ne nous voilons pas la face, la France a un rôle prépondérant à jouer. À quand une décision courageuse concernant le lancement de ces projets et le choix des sites retenus ?

l'étude des options technologiques qui pourraient assurer la fermeture complète du cycle sur le long terme. Jusqu'à présent, les efforts de recherche se sont concentrés sur le déploiement de la filière des réacteurs à neutrons rapides de quatrième génération refroidis au sodium. Pour autant, le constat partagé par le Gouvernement et la filière est que les ressources en uranium sont abondantes et disponibles à bas prix au moins jusqu'à la deuxième moitié du XXIsiècle. Dans ces conditions, le déploiement de réacteurs à neutrons rapides n'apparaît pas nécessaire avant cet horizon. C'est ce qui a conduit le Gouvernement à réorienter les efforts de R&D vers un programme visant à renforcer et à maintenir les compétences sur la connaissance de la physique des réacteurs à neutrons rapides et des procédés du cycle associés. S'agissant des programmes EPR, il est prévu d'étudier tous les scénarios dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, depuis

la question de la démonstration par la filière de sa capacité à relever, sur le plan de la qualité industrielle et de la maîtrise des délais et des coûts, le défi que représenterait la construction de réacteurs est bien sûr primordiale.

Il y a maintenant plus de soixante-quinze ans, la France décidait de canaliser la puissance de l'eau par la construction de barrages, afin d'en prendre le meilleur et de créer de l'énergie. Aujourd'hui, d'aucuns verraient bien ces chefs-d'oeuvre nationaux concédés à des puissances économiques étrangères.

Notre pays serait donc le premier à ouvrir ce secteur à la concurrence. En 2016, lors de la transposition de la directive européenne qui prévoit l'ouverture des concessions de service public à la concurrence mondiale, la France n'a pas prévu d'exempter ses barrages, à l'inverse d'autres pays européens. La gestion de nos installations hydroélectriques est ainsi à la merci des intérêts de puissances étrangères et d'acteurs privés. Les bénéfices estimés à environ 1,25 milliard d'euros viennent logiquement attiser la convoitise des investisseurs privés. Par ailleurs, comme le pointe un rapport de 2013, une hausse mécanique du prix de l'électricité pour les consommateurs serait inéluctable. N'avons-nous pas déjà vécu cela lors de la privatisation des autoroutes ? N'est-ce pas suffisant ? Les Alpes comprennent pas moins de 132 barrages, dont 26 en Savoie. Un large consensus se dessine dans la population, comme chez les élus locaux et nationaux, pour rejeter cette mise en concurrence jugée Comment pourrait-on sacrifier un tel patrimoine, source d'emplois qualifiés, directs, indirects et induits pour des femmes et des hommes dotés d'un haut niveau d'expertise ?

de concessions. Le droit français, en conformité avec le droit européen, prévoit par ailleurs que les concessions hydroélectriques échues doivent être renouvelées par mise en concurrence. Ce sujet préoccupe les gouvernements successifs depuis un certain temps,

aux concessions dans le cadre d'une société d'économie mixte hydroélectrique, à la possibilité de regrouper des concessions hydrauliquement liées pour faciliter leur exploitation et favoriser la sûreté, à l'existence d'un mécanisme de prolongation contre travaux dans le respect de la directive Concessions et, bien entendu, à la préservation du statut des personnels

mettre en place un opérateur qui pourrait être public à 100 % et qui, de ce fait, pourrait échapper à la mise en concession. Voilà les différentes pistes sur lesquelles nous travaillons actuellement.

La vision stratégique de long terme sous-tend l'ensemble du dossier de la politique énergétique. Si les choix s'opèrent dans l'instantanéité d'un seuil de rentabilité économique, cela signifie que les enjeux environnementaux sont secondaires, ce qui n'est pas acceptable dans un contexte d'urgence climatique. Les consommations individuelles, les mobilités, les pratiques de la société en général doivent se verdir et se décarboner, mais encore faudrait-il savoir comment. En effet, comment inciter le consommateur à acheter des véhicules électriques si l'électricité provient d'une centrale à charbon ou d'une source polluante ? Si l'on veut gagner, il faut que les choix soient lisibles. On ne peut pas bâtir une incohérences, le risque premier étant de perdre le consommateur en chemin. Or c'est lui, en grande partie, qui est la clé. Le président Marseille l'a très justement rappelé, l'exemple de la filière nucléaire Celle-ci fut par le passé un choix stratégique fort, permettant une production décarbonée dont nous avons la maîtrise. Cependant, force est de constater que, déjà à l'époque, les visions stratégiques furent incomplètes et partielles, puisque l'épineuse question du traitement des déchets fut un peu « zappée ». À La Hague, nous voyons aujourd'hui des files d'attente de déchets, qui imposent des solutions de stockage d'urgence. On ne peut pas travailler comme cela. À la croisée des chemins, au moment où les mobilités électriques vont entraîner des hausses de consommation, où le parc vieillit, où l'EPR a plombé les comptes, la France n'a pas les moyens de ses hésitations. Le choix d'un mix énergétique cohérent doit se faire sur des bases stables et dans la durée. Pourtant, la PPE est encore en débat ! Son acceptabilité est indispensable, c'est une question de crédibilité. On ne doit pas voir fleurir des projets éoliens déconnectés de la carte des vents. Vous nous avez rassurés sur le fait que vous comptiez exploiter au maximum les ressources hydrauliques, l'hydroélectricité étant à ce jour la seule énergie réellement renouvelable, flexible et non polluante. Vous avez entendu sur ce sujet combien les attentes des territoires On ne peut se priver de faire une place à l'autoproduction, la ressource de proximité étant forcément la meilleure. On ne peut déconnecter les politiques tarifaires et fiscales des politiques environnementales. Il faut se donner les moyens financiers de la transition. On ne peut décider de baisser la part du nucléaire sans savoir comment la compenser. On ne peut pas demander au secteur de l'industrie électrique de faire les frais, en maintenant l'équilibre de son modèle économique, de nos incohérences et de nos changements de cap. On ne peut placer les agents d'EDF dans des situations incertaines et préjudiciables. Il faut au contraire donner aux grandes compagnies d'électricité, dans un contexte où l'évolution technologique est fulgurante, les moyens de conserver l'équilibre dans la durée. De la stabilité du système dépend aussi la sécurité d'approvisionnement. L'arrivée d'énergies renouvelables intermittentes, rémunérées avec des garanties spécifiques, a bousculé de manière significative les fournisseurs d'électricité européens. Ceux-ci ont été obligés de se restructurer et de redéfinir leurs stratégies. Des changements structurels s'opèrent en amont, de nouveaux entrants arrivent sur le marché de l'énergie, y compris les autoconsommateurs. À l'autre bout de la chaîne, du côté des utilisateurs, on observe également des changements profonds, largement influencés par les politiques publiques, ce qui permet de souligner une nouvelle fois l'indispensable cohérence entre l'amont et l'aval, entre la production et l'utilisation, entre la composition du mix et le travail auprès des consommateurs et, entre les deux, la position stratégique des réseaux. De nouveaux services sont devenus nécessaires, comme la flexibilité, l'aide au contrôle de la consommation, dans un univers énergétique devenu intelligent. Le numérique, en contribuant en amont à lisser les apports dans le réseau de productions intermittentes et en répondant aux attentes des consommateurs en aval, sera une aide précieuse pour conserver l'efficience économique du système. La digitalisation doit permettre au client de devenir réactif aux changements de prix, ce qui constitue peut-être un levier pour aller vers une tarification plus environnementale. Le paquet énergie propre- vous en avez parlé -, qui a été adopté au printemps par l'Union européenne, comporte plusieurs mesures susceptibles d'accélérer la reconfiguration du secteur. Il existe donc des pistes dans ce contexte en évolution permanente. EDF peut s'adapter, à condition que l'on fasse ce choix et qu'on lui en donne les moyens financiers. Vous nous avez dit, madame la ministre, que nous savons où nous voulons aller. Reste maintenant à savoir avec qui : est-ce avec Hercule ? Est-ce avec Astrid ? Est-ce, oui ou non, avec EDF ? Nous en avons terminé J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est parvenue à l'adoption d'un texte commun.